La séance est ouvert. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, nous n'avons pas reçu d'observation.

J'ai consulté le sénat du regard. Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Alors revue jour après les questions d'actualité au gouvernement, la séance est retransmise en Direct sur France 3 sur Public Sénat sur le site internet du Sénat et sur Facebook, chacun sera attentif à 2 choses : une évidente : le respect des uns des autres une seconde qui nécessite un peu de volonté, le respect du temps à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, monsieur le président, Mesdames, messieurs, ministre monsieur le 1er ministre ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre la situation des djihadistes de retour sur le territoire national et européen constitue une cause d'inquiétude à Brest moyen et et et long terme, nous les avons pas vraiment vu partir, j'ai quelques doutes sur le fait que nous, les repères rayons quand ils reviennent, les femmes présentant un danger à peu près équivalent aux hommes quant aux enfants, leur prise en charge doit être assuré en fonction de l'orage, compte tenu des traumatismes vécus plusieurs traumatologie évoque un fort potentiel de dangerosité, à terme, nous le savons, à ce stade, aucune politique de des radicalisation ne semble convaincante, ni en France ni à l'étranger et pourtant, nous ne pourrons pas nous contenter Nicolas Roch ni forum ni de rapports, les détentions ne seront pas éternelles aussi Monsieur le 1er ministre ma question est extrêmement simple : quels éléments concrets, avez-vous aujourd'hui et pouvez-vous nous donner pour répondre à notre inquiétude comment faisons-nous avec ces djihadistes de retour sur le territoire national, je vous remercie. Pour vous répondent : la parole et faire Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Monsieur Collomb la parole. Monsieur le président, mais dames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet. Vous le savez le gouvernement porte une attention particulière aux problèmes des retournés. Les accords qui ont été passés entre la Turquie et la France, dit accord nous permettent d'avoir un regard particulièrement attentif sur celles et ceux qui reviennent des théâtres de guerre syro-irakien actuellement, ce sont plus de 240 majeur et plus de 50 mineurs dont la plupart ont moins de 12 ans qui sont revenus depuis 2012 sur le sol français, vous le savez sans doute, le principe d'un traitement judiciaire et systématique, retenons une qualification de nature criminelle et le procureur de la République de Paris et celui qui a la charge de cette question, la prise en charge des retourner se fait donc depuis 2015 par un placement systématique en garde à vue, des femmes et des hommes majeurs et des quelques mineurs combattants après leur placement en garde à vue, le juge des libertés et de la détention peut décider d'une incarcération et une très grande majorité de retenue est actuellement en prison plus de 130 les les autres, ceux qui sont en liberté, ils sont tous évidemment l'objet d'un suivi administratif par les services de renseignement DGSI RT soit d'un suivi judiciaire lorsque les juges ont décidé d'un placement sous contrôle judiciaire, ainsi ce problème est parfaitement prise en charge aujourd'hui. Qui monsieur Madame Goulet. Monsieur le ministre, gêne 2 pas de votre de votre bonne foi, ni de la bonne foi de ce gouvernement qui a été aussi la bonne foi du gouvernement précédent, et de l'ensemble du Parlement qui a largement soutenu les dispositions qui ont été votées depuis 2 ans, voire 3, je voudrais simplement vous dire que Frontex fonctionne mal que il y a un il faut des moyens en hommes, il faut des moyens en matériels, il faut des moyens de contrôle de passeport, il faut des moyens de contrôle de frontières, franchement je je je ne partage pas votre votre position et je pense qu'il faut être encore beaucoup plus, beaucoup plus vigilant, et en tous les cas, accorder à ce à ce sujet une attention majeure, et notamment au niveau au niveau européen, nous, nous ne pourrons pas en sortir autrement qu'en confortant nos frontières, je vous remercie. La parole est au président François Patriat pour le groupe, la République en marche, vous avez la parole monsieur le président. Merci monsieur le président. Monsieur le 1er ministre lundi dernier à l'issue d'une très longue journée de concertation Les ministres des Affaires sociales de l'Europe. Ont abouti à compromis historique sur la révision de la directive des travailleurs détachés, c'est la. C'est là une avancée importante qui répond aux voeux du président de la République qui avait voulu que nous modifions le cadre juridique pour les travailleurs détachés de façon arriver à l'Europe qui protège, c'est à l'issue d'un long tour des capitales européennes, que le chef de l'État a réussi à convaincre ceux qui étaient réticents jusqu'à présent, aboutissant en cela au fait que demain, il y avait dans notre territoire, il a beau jeu d'autres territoires, des gens qui profitait des différences, protection sociale et salariale qui était de 1 à 3 dans l'Europe à 15 et qui sont dans l'à 10 dans l'Europe à 28, vous comprendrez que les travailleurs ce tronçon en tirant un peu mieux protéger les entreprises subiront moins la concurrence internationale et nous aboutissons ainsi à 4 avancées majeures la 1ère c'est que les salariés dans tous les pays d'Europe seront payés au tarif mais chaque pays d'Europe, la 2ème avancée c'est que la fraude sera aujourd'hui mieux contrôlés, la 3ème, c'est que la durée de travail du travailleur détaché n'excédera pas maintenant 12 mois au lieu de 2 ans et plus, aujourd'hui, et en 3ème lieu dans le domaine routier, la voie est ouverte maintenant puisqu'ils relèveront de la directive à ce qui est des améliorations dans les 6 mois qui viennent, ma question, monsieur le 1er ministre comment voyez-vous maintenant la suite de décisions historiques que j'espère me chers collègues, vous êtes tout ça lui avec moi merci. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Patriat merci de vos propos qui viennent saluer un investissement l'investissement du du président de la République, c'est vrai, l'avait 6 membres du gouvernement de l'ensemble de la diplomatie française, mais je voudrais si vous me le permettez, notez et remercier le travail exceptionnel fait à la fois par l'Muriel Pénicaud, madame la ministre du Travail et par Nathalie Loiseau, ministre de l'Europe, qui ont toutes les 2 de façon incessante parcourent les capitales européennes pour expliquer et convaincre du bien-fondé de la position française. Si nous revenons un peu en arrière, mesdames et messieurs les sénateurs. Personne ici, je crois ne il y a 3 ans. Que la situation qui prévalait sous l'empire de la directive telle qu'elle existait à l'époque était une bonne situation, je n'ai jamais vu aucun parlementaire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, se lever pour dire il y a 3 ans sa directive vraiment aller parfaite surtout la chanson pas donc la solution n'était pas satisfaisante, il y a un peu plus d'un an, lorsque la Commission européenne a déposé sur la table sa proposition, peu de gens, imaginez qu'serait susceptible de rencontrer rapidement un accord parce que de très nombreux pays, disait qu'il ne voulait pas d'une modification de la directive sur les travailleurs détachés lundi dernier après un travail de conviction très important après que nos partenaires les plus proches. Eurent décidé de se rallier à nous et que d'autres partenaires plus lointain, je pense à un certain nombre de pays qui se trouve à l'Est de l'Europe que l'on n'attendait pas forcément sur ce sujet et décidé de nous rejoindre, nous avons obtenu un accord j'ai la conviction et c'est une conviction largement partagée que l'accord que nous avons obtenues sur la directive travailleurs détachés. Provoque une situation qui est bien meilleure aujourd'hui qu'elle n'était hier.

et encore beaucoup de travail pour faire en sorte que les éléments soient complètement stabilisée car. La commission emploi du Parlement européen a pris une position il y a quelque temps qui n'est pas identique à celles prises par les États membres lundi soir qu'il n'est pas non plus très éloigné, mais la commission emploi après qu'un travail très intéressant, a été réalisée par notre compatriote Élisabeth Morin Chartier a pris une position qui me paraît pouvoir être rapproché de façon rapide grâce à dialogue ou, plus exactement. Un trilogue entre la Commission, les États membres et les parlementaires du Parlement européen. je souhaite que cette discussion s'engage dès que possible car. Pour l'ensemble des pays. Des États pour l'ensemble des travailleurs européens, pas simplement les travailleurs français pour l'ensemble des travailleurs européens, ce texte représente une protection supplémentaire il importe donc qu'il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible, et que donc les discussions entre les acteurs encore autour de la table, puisse avoir lieu dans les plus brefs délais un mot pour dire que l'accord auquel nous sommes parvenus, lundi soir, indique que la directive s'applique aux travailleurs du secteur des transports la rappelle qu'elle s'applique aux travailleurs des transports compte tenu des spécificités évidente de ce secteur des discussions interviendront pour préciser les conditions dans lesquelles les contrôles, notamment, s'applique au aux travailleurs qui sont par nature mobile quand il s'agit de du secteur des transports, c'est donc une discussion qui est devant nous et qui devra intervenir un pigment. Je dois dire, Monsieur le Président pour conclure que le travail qui a été effectué est un travail de constitution d'une majorité européenne, c'est un travail qui s'adresse à tous les partenaires de la France, pas simplement aux partenaires les plus traditionnels et les plus importants par leur nombre, par leur influence à tous les partenaires de la France, ce qui a prévalu 7 donc une méthode nous affichons clairement nos ambitions et nous les disons clairement : nous essayons de constituer des majorités avec un travail très fin, auprès de l'ensemble de nos partenaires, nous ne jouerons pas l'opposition, qui est une opposition mortifère pour l'Union européenne entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, c'est un point sur lequel je vais insister dans la discussion qui est intervenu, lundi soir, l'ensemble des pays à veiller à ce que cette opposition ne prévalent pas et à ce que des pays qui sont situés à l'Est puisse rejoindre le compromis c'était précieux pour l'avenir de ce texte et c'est à mon avis précieux pour le reste de l'Europe. La parole est maintenant notre collègue Raymond Vall pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, monsieur le président. Merci monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire monsieur Nicolas Hulot en 2014, le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mère décide de lancer le programme territoire énergie positive pour la croissance verte afin de territorialiser la politique de transition énergétique 554 territoires sont labellisés sur l'ensemble du territoire métropolitain d'outre-mer, ce qui représente 15000 communes et concerne près de 40 millions d'habitants, le bilan fait en avril 2017 est très positif puisque l'effet de levier obtenus par le fonds permet de multiplier par 3 les investissements des collectivités avec des résultats concrets pour l'environnement, l'économie locale et l'emploi, à savoir économie de 800 10000 tonnes de CO 2 plus d'un 1000000 4 de foyers supplémentaires alimenter aller avec des énergies renouvelables, plus de 3500 véhicules électriques et hybrides 4 millions de mètres carrés de surface photovoltaïque déployés et 200 territoire 0 pesticide alors Monsieur le Ministre, vous comprendrez bien que votre circulaire du 26 septembre dernier accompagné le 5 octobre suivant Dundee de d'interprétations qui ont pour but d'arrêter tous les projets possibles afin de limiter le montant des crédits de paiement à 400 millions d'euros, alors que les engagements conclus s'élève à plus de 750 millions d'euros, a déclenché un véritable tremblement de terre au sein de ces territoires qui, eux, se sont engagés, fort de la signature de l'État auprès de leurs populations et parfois des entreprises locales, monsieur le ministre s'était dit scission brutale et perçue comme injuste et doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation plus précise avant qu'elles viennent alimenter une une fois encore le sentiment que la parole de l'État n'est plus respecté. Vous répondent : la parole Corinne Istres d'État, ministre de la transition écologique et solidaire monsieur Hulot. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Val. Vous imaginez bien que ça n'est pas de gaieté de coeur que j'ai déclenché cette onde sismique je partage comme vous la conviction et vous en avait fait la démonstration que la transition écologique passe par les territoires territoires effectivement dans la dynamique de la loi de la transition énergétique de 2015 et, à l'appel de l'État, vous l'avez mentionné des milliers de collectivités se sont engagées dans des projets transition qu'en se regroupant entre elles, effectivement, en associant des acteurs économiques locaux les collectivités, les collectivités françaises sont en pointe dans la lutte contre le changement climatique pour accompagner cette dynamique, une enveloppe spéciale de transition énergétique a été mise en place, mais elle n'a été toutefois été financés qu'en 2015 et en 2016 à hauteur de 400 millions d'euros de crédits de paiement, le problème que j'ai découvert avec les conventions conclues avec les collectivités locales et territoire représente un total de 748 millions d'euros, c'est au regard de cette insuffisance de crédit que j'ai effectivement adressé une directive aux préfets de région le 26 septembre dernier pour trouver la solution, j'ai besoin d'abord d'un état des lieux précis on doit mesurer le niveau d'avancement des projets et identifier ce qui rencontre des difficultés de mise en oeuvre afin de préciser le niveau d'engagement financier de l'État, la collecte d'informations est en cours et il est donc trop tôt pour répondre à toutes les interrogations qui nous remontent, mais je sais qu'il faut de la confiance entre l'État et ses territoires, donc je peux vous rassurer sur le fait que la parole de l'État sera tenu les projets déjà lancés, qui seront menées à leur terme dans les délais seront financées, donc nous allons continuer à travailler dans le cas de la conférence nationale des territoires car les territoires Jean convaincu comme vous sont la clef pour réussir ma propre transition écologique. Merci. Quelques secondes, merci Monsieur le président, Monsieur le ministre, j'ai bien enregistrer ce que vous avez dit je voudrais simplement vous dire très sincèrement, si vous voulez pouvoir compter sur ces territoires, pour mettre un à votre plan climat très ambitieux que vous avez présenté en 2017, ne laissez pas tomber, il compte sur vous. Si la parole est à notre collègue Christine Pruneau pour le groupe. Communistes, républicains, citoyens et écologiste pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Monsieur le Président ma question était adressé à monsieur le ministre des Affaires étrangères doc, madame la ministre, après avoir déjà passé 7 ans en prison, notre compatriote Salah Hamouri a été une nouvelle fois arrêté par la mi-israélienne le 23 août dernier ce 18 septembre un tribunal militaire l'a de nouveau condamné à une détention administrative, détention, vous le savez, qui peut-être nous valable à l'infini, sans plus de justification, ses avocats n'ont toujours pas pu prendre connaissance des preuves sur lesquels ces incriminations se fonde sa famille n'a toujours pas pu lui rendre visite, parchemin un acharnement politique contre un défenseur des droits humains, dont le dossier est vide face aux méthodes israéliennes arbitraire et sur bien des points contraires au droit international, le Quai d'Orsay a enfin dénoncé hier cette détention administrative, il était temps, il était temps que notre pays interviennent en faveur de l'un de ses ressortissants, victime d'une injustice le légitime combat de Salah Hamouri pour la Palestine pacifique, il ne ressemble en rien à une entreprise terroriste, madame la ministre, être préoccupé et dénoncer c'est bien, mais l'exigence d'une libération immédiate de Salah Hamouri demeure : que comptez-vous faire. Madame Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes avaient la parole, Madame la Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice pruneaux, le gouvernement partage votre préoccupation sur la situation de Salah Hamouri ressortissant palestinien, mais aussi français et donc notre camp patriote comme vous l'avez dit, il a été arrêté le 23 août dernier le juge de District israélien a confirmé le 18 septembre sa détention administrative, la dernière audience en appel à l'encontre de cette décision de mise en détention, ses tenues à la Cour suprême israélienne de Jérusalem, le 22 octobre ni notre compatriote ni ses avocats n'ont pu avoir connaissance des charges retenues contre lui. Comme tous les Français détenus à travers le monde Salah Hamouri bénéficie pleinement de la protection consulaire française en conformité avec la Convention de Vienne, notre consul général va rendu visite sur son site de détention et le consulat général est présent à chacune des audiences publiques auxquelles il a comparu, nous avons fait part aux autorités israéliennes de toute l'attention que nous portons à son cas et de notre préoccupation face à l'usage extensif de la détention administrative, je le rappelle, lui, l'utilisation abusive et systématique de la détention administrative porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, nous demandons que l'ensemble des droits de notre compatriote soit respectée et nous espérons sa libération, nous sommes aussi intervenus afin que de demander que sa famille puisse y rendre visite soyez assurée, Madame la sénatrice de l'attention avec laquelle nous allons continuer à suivre la situation de monsieur Hamouri et pas seulement par des déclarations publiques merci. Merci, non Bruno. J'ai pris bonne note, Madame la Ministre de l'attention que que vous portez à à cette affaire, vous avez su engager enfin au niveau des autorités des dossiers similaires ce que vous avez pu exiger de la Turquie, qu'il n'est pas non plus un pays démocratique pour la libération de loup bureau nous souhaiterions que vous ayez la même volonté et exigences bien sûr puisque ni l'un et l'autre n'étaient des terroristes en ce que nous voulons, nous, ce n'est, c'est la libération immédiate, pas dans 2 mois pendant 3 mois, pendant 6 mois, c'est vraiment une volonté de beaucoup ici sur nos banques et au niveau associatif, je vous remercie de bien vouloir être encore plus exigeants, le ministre. La parole est maintenant notre collègue Bernard Jomier pour le groupe socialiste et républicain, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des solidarités, de la santé en 2016 plus d'un quart des assurés sociaux ont renoncé à des soins si les causes de ce renoncement sont multiples : tous les spécialistes de la question sont unanimes pour affirmer que l'extension des dispense d'avance de frais est un levier d'action majeure pour résorber ce problème, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie l'a encore rappelé hier, lors de son audition devant notre commission des affaires sociales, alors que le vote de la loi de modernisation de notre système de santé avait marqué un acte décisif en ce sens, vous récentes déclarations entretiennent le flou et nous font craindre un retour en arrière, pourquoi insinuer le doute sur une mesure qui fonctionne et s'applique déjà, comme le souligne le rapport de l'IGAS d'octobre 2017 sur le terrain au quotidien le tiers payant et mis en place par les professionnels de santé pour les patients pris en charge à 100 pourcent par par la Sécurité sociale, il reste oui à résoudre des difficultés techniques sur la part complémentaire pour aboutir à un système qui doit bien sûr être simple et affluent unique pour les professionnels de santé, je tiens à rappeler qu'en Europe, 24 pays sur 28 pratique d'ores et déjà la dispense totale de paiement en annonçant la généralisation du tiers payant, nous avons créé une forte attente une approbation massive des assurés sociaux, nous devons nous montrer à la hauteur de ces attentes et poursuivent l'action engagée en faveur de la liste pense de paiement et dans le respect de la loi monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous confirmer l'engagement pris par le président de la République dans la mise en place de cette mesure, pouvez-vous nous éclairer sur le délai dans lequel les Français pourront bénéficier d'une dispense complète d'avance de frais pour les actes pris en charge par l'assurance maladie, je vous remercie. monsieur Christophe questionnaire. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Jomier. Comme chacun d'entre nous, nous sommes attachés à l'accessibilité aux soins, la plus large possible, jamais, jamais, l'argent ne doit être un obstacle pour faire en sorte que telle ou telle personne ne puisse en bénéficier, on voit bien depuis quelques années, la montée en puissance de dispositif assez similaire à celle de la généralisation du tiers Pierre, on le voit en particulier pour l'ensemble des publics qui sont en situation de précarité, notamment les bénéficiaires de la CMU complémentaire, mais aussi ceux qui étaient dans l'aide d'une complémentaire santé ou enfin ceux qui souffrent d'une ALD d'une affection de longue durée, nous y sommes tous attachés, mais au fond, dans ce pays on se complaît trop souvent à confondre les droits réels et les droits formels, il nous arrive dans nos assemblées de penser qu'il suffit de voter un texte pour garantir sa mise en avant, or, la réalité est un petit peu plus complexes, et la ministre que j'esquisse mélo bon sur le PLFSS à l'Assemblée nationale a immédiatement légendes, c'est une mission d'inspection de l'IGAS pour faire un point sur la faisabilité de la mise en oeuvre dans de bonnes conditions pour ne pas fragiliser les médecins qui sont aujourd'hui déjà dans une difficulté que chacun, chacune d'entre nous connaissons et pour faire en sorte effectivement que nous ne reculerons pas pour celles et ceux qui ont besoin de la généralisation de ce dispositif et donc l'engagement que nous avons pris, c'est d'abord de prendre acte, acte de l'impossibilité technique de respecter les délais sous peine de fragiliser l'ensemble de l'offre de soins sur le territoire mais de fixer l'ambition cette ambition, c'est de faire en sorte que le tiers payant soit généralisable le plus vite possible qu'il soit garanti pour toutes celles et tous ceux qui en ont le plus besoin immédiatement et qui soit généralisable pour toutes celles sous ceux qui sont en lien avec leur médecin en capacité de le mettre en avant la ministre vous présentera dans quelques jours, dans quelques semaines, le plan d'action que nous voulons mettre en oeuvre et nous voulons faire en sorte que cet objectif se traduise dans les faits concrets et pas seulement dans les déclarations d'intention, je vous remercie. Merci Monsieur le secrétaire d'État, mais je ne peux pas croire que en France au XXIe siècle des problèmes informatiques indique pas si complexe que ça pu mettre à bas une avancée sociale fort merci.

Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, à compter du 1er novembre les officiers d'état civil seront chargés de toute la procédure du pacte civil de solidarité déclaration conjointe des partenaires modification et dissolution de la convention du Pacs, publicité, réalisation de statistiques semestrielles, l'objectif que l'on ne ne peut qu'approuver est avant tout d'alléger la charge des tribunaux pour les recentrer vers des missions purement juridictionnel, c'est également une mesure de simplification au bénéfice des citoyens qui ne seront plus contraints de se rendre au tribunal, enfin cette mesure rejoint la pratique de la majorité des pays européens, on peut également saluer ce transfert qui peut apparaître comme une reconnaissance de la commune et de ses élus qui constituent le maillage démocratique de tout notre pays, pourtant, il reste à quelques jours du transfert une ombre au tableau : la compensation financière de l'État, au-delà du fait que ce changement imminents n'est pas encore tout à fait prêt dans un grand nombre de communes, ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter à la gestion des passeports biométriques des cartes d'identité du changement de prénom du Duce, du système commode avec de plus, la loi stipule que 284 communes auront à traiter les données numériques et les dossiers papier Despax détenu par les greffes des tribunaux d'instance et de grande instance, et ce pour tous les justiciables des communes de leur ressort, il va donc souvent falloir aménager des locaux restructuré des services donc des dépenses supplémentaires pour les communes, je vous demande donc, Monsieur le Ministre quelles compensations seront dégagés pour que ce nouveau transfert de charge ne viennent pas alourdir les Budgets communaux malmené ces dernières années. On vous répond : la parole est à Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur s'est mise d'État. Mesdames, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices madame la sénatrice. Vous attirer mon attention sur 2 questions. La première. Concerne le transfert de gestion. De demandes de passeport excusez-moi. Qui a déjà été réalisé. Je vous rappelle que c'est une question ancienne. Vous parlez des changements de prénom. C'est aussi une question ancienne, enfin vous m'interrogez sur le Pacs qui a été effectivement transférés en mairie par la loi de justice 21ème siècle en novembre 2016. Vous estimez qu'il aurait été nécessaire de prévoir une compensation financière pour cette nouvelle attribution. Cette question a été tranchée à l'occasion de la loi Justice 21ième siècle par une décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a décidé, je cite : l'obligation pour l'État de compenser financièrement l'exercice de certaines compétences, mais ceci ne s'applique pas à celles qui sont exercées au nom de l'État, or le Pacs est une mission exercée au nom de l'État. Malgré cette jurisprudence nous avons inscrit aujourd'hui 22 millions d'euros de crédits, donc j'aurai l'occasion de vous parler, mais le Conseil constitutionnel a ajouté que, s'agissant du Pacs dans les mêmes décisions, il dit que le montant des sommes en jeu n'est pas telle qu'il porte atteinte à la libre administration des communes concernées. Monsieur le ministre, je souhaiterais toutefois que vous puissiez examiner la possibilité pour les 284 communes qui devront assurer un service public pour des non-résidents, insiste d'obtenir non pas une compensation mais une indemnisation spécifique, comme ce fut le cas pour l'instruction des passeports biométriques, je vous en remercie. La parole est maintenant Madame Dominique Estrosi Sassone pour le groupe, les républicains. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la cohésion des territoires depuis l'annonce brutale d'une baisse de 5 euros par mois des APL au cours de l'été, le gouvernement continue de s'enfoncer dans sa stratégie logement au travers de mesures injustes à l'emporte-pièce, dictée par la seule volonté de réaliser 1,7 milliards d'euros d'économies dans le budget 2018, la baisse de 60 euros par mois des APL, avec pour contrepartie la baisse des loyers équivalente imposée aux organismes HLM et mortifère pour le logement locatif social pour l'accession sociale et injuste pour nos concitoyens les plus modestes, ce sont 2,2 milliards d'euros d'autofinancement qui ne seront plus réinvestis dans la production neuve dans la réhabilitation dans l'entretien et la réparation du parc existant, les contreparties financières telles qu'elles sont proposées aujourd'hui ne sont pas entendable parce qu'elles ne produiront un tant soit peu des effets significatifs qu'à moyen et à long terme cette réforme Monsieur le Ministre, telle qu'elle est arrêtée aujourd'hui fait que des perdants, les locataires qui n'auront pas de pouvoir d'achat augmenter et qui verront leurs conditions d'habitat se dégrader, les collectivités locales qui garantissent des emprunts des organismes dont 100 à 200 devraient être en faillite, le renouvellement, le programme de renouvellement urbain, qui devraient être impactés et enfin l'ensemble de la filière du secteur du bâtiment qui va voir ses commandes chuter alors Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt à revoir votre copie à prendre des mesures susceptibles de ne pas obérer l'avenir d'un secteur essentiel pour la solidarité nationale, l'emploi et l'aménagement du territoire. du territoire. Puis au secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion sociale. Monsieur de Normandie. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, madame la sénatrice je connais et je salue votre engagement sur la politique de logement, et notamment sur la rénovation urbaine à Nice pour laquelle vous êtes au combien engagé depuis des années, quelle est la réforme que nous souhaitons pour le logement social. On part d'un constat aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 4 millions et demi de logements sociaux en France et il y a un 1000000 et demi de nos de nos concitoyens de ménages qui sont en attente d'un logement social, donc le constat c'est que des facteurs, aujourd'hui il n'y a pas assez de logements sociaux en France dans notre pays qu'est-ce qu'on fait discute dont on discute avec l'ensemble des bailleurs sociaux, elle repose sur plusieurs piliers : un 1er pilier qui est la mobilité au sein du Parti social, c'est-à-dire pouvoir révisé tous les 6 ans, les situations des uns et des autres, vivant dans les logements sociaux pour pouvoir permettre d'améliorer cette mobilité, le 2ème, c'est de pousser un regroupement des bailleurs sociaux pour avoir des bailleurs sociaux, plus fort, capable d'accueillir plus de politique de public fragile et capable également de faire plus d'investissements, le 3ème pilier de s'être réforme c'est de faire plus d'accession sociale en cédant plus de logements par les bailleurs sociaux qui rapporte plus de capacité d'autofinancement pour ces derniers, et le 4ème volet que vous mentionnez dans votre question, c'est d'améliorer les conditions de financement de l'ensemble de ses bailleurs sociaux car c'est nous qui les finançons améliorer ses capacités de financement, c'est de faire des prêts de plus longue devrait essayer d'apporter des capitaux, c'est de donner 3 milliards d'euros pour faire de l'efficacité énergétique et diminuer les charges et, en contrepartie de ça, c'est avec les bailleurs sociaux, lutter contre la spirale infernale infernal d'os des appels, et donc nous discutons, je dois dire tous les jours avec l'ensemble de ses bailleurs sociaux avec le 1er ministre avec chaque maison, les bailleurs sociaux eux-mêmes que nous avons revu encore ce matin,

cette concertation elle continue et cette concertation, nous avons bon espoir de la terminer dans les tous prochains jours avec une encore congrès on va temps le bénéfice pour les locataires qui ne seront pas impactés, je vous remercie. Madame Estrosi ça sonne. Que le dialogue continue, personne ne va s'en plaindre, Monsieur le Ministre, seulement à cette injustice profonde par cette réforme des APL vous commettez un contresens économique terribles, parce que ce contresens économique traduira que la charte de l'offre fera pschitt et j'ai bien entendu le président de la République, dire qu'il se basait surtout avant tout sur des mesures qui soient pour relancer l'offre de logements et donc là au contraire vous obérer le choc de l'offre et si vous voulez conduire vraiment conclure, logement, il faut que des réformes soient profonde, structurelle et que ne soient pas des coups de rabot des variables d'ajustement assez la parole est à notre collègue Laurent Lafon. Pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Ministre d'État, le Grand Paris Express avec ses 200 kilomètres de lignes automatiques et ses 68 nouvelles gares est un projet structurant permettant enfin d'améliorer le quotidien et le cadre de vider de nombreux franciliens, il constitue également pour les territoires et les communes qui bénéficieront d'une des gares un puissant levier de développement économique et de construction de logements, le gouvernement a demandé pendant l'été, de procéder à une actualisation du coût du projet, il apparaît désormais que évaluée à l'origine à 25 milliards d'euros le coût du projet serait dans une fourchette basse à 28 milliards et dans une fourchette haute, à 35 milliards ce surcoût suscite de nombreuses inquiétudes chez les élus locaux, dans le Val-de-Marne en Essonne et en Seine Saint-Denis notamment élu qui s'interroge sur l'origine de ces dépassements budgétaires et les financements qu'il sera nécessaire de trouver désormais mais aussi sur le respect du calendrier et l'engagement que leur projet sera bien réalisé dans sa totalité, alors que la mise en oeuvre du nouveau réseau est officiellement prévue entre 2000 22 et 2030, il est nécessaire aujourd'hui de répondre aux interrogations et aux inquiétudes par des réponses claires et précises, aussi Monsieur le Ministre d'État, ma question est simple : l'apparition de ces surcoûts va-t-elle amener l'État à remettre en cause la réalisation de ce projet dans sa globalité à à modifier le calendrier prévu à l'origine à réétudier le financement et la participation des différents acteurs. Bonjour et prendre la parole est à madame brune Poirson, secrétaire d'État. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs Monsieur sénateur Laurent Lafon je tiens tout d'abord excusez Élisabeth Banks qui a pas pu être présent aujourd'hui parce qu'elle est à Belfort avec Bruno Le Maire et d'emblée, je veux rappeler l'importance du projet du Grand Paris Express qui permet de faciliter la mobilité quotidienne de tous les Franciliens, en privilégiant les déplacements qui contournent Paris, c'est un projet qui redessine véritablement la géographie, l'Île-de-France, en réduisant l'opposition entre Paris et sa banlieue, ce projet, il n'y a absolument indispensable pour maintenir l'Île-de-France dans les tout premiers rangs des métropoles mondiales et je veux vraiment insister sur le fait que le schéma d'ensemble n'est pas remis en cause, il est sanctuarisé. Mais il faut que nous donnions compte de 2 éléments nouveaux : d'abord la perspective des eaux implique en 2024 et puis aussi les surcoûts très importants qui sont apparues au cours des 3 dernières années, et c'est pour ça que le préfet de région a été chargé de faire un point précis sur le programme de réalisation du Grand Paris Express et le préfet a remis son rapport au 1er ministre à la fin du mois de septembre, ces propositions sont actuellement en cours d'analyse et le gouvernement annoncera chez soi très prochainement avec la volonté réaffirmée de préserver au mieux les objectifs de ce projet qui, je répète, est absolument essentielle pour l'Île-de-France.

au regard de votre remarque sur les Jeux olympiques, je ne voudrais pas et nous sommes nombreux dans ce cas-là, à ce que les Jeux olympiques, aboutissent à une priorité nisation du réseau pour les sites qui seront desservies, laissant les autres territoires qui eux ne bénéficieront pas de sites olympiques prendre du retard en terme de transport en commun. Merci, la parole est maintenant notre collègue. Didier Rambaud pour le groupe, la République en marche. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État au numérique concerne plus particulièrement le sujet de la taxation des géants de l'internet, ces fameux GAFA aujourd'hui, il est facile aux entreprises du numérique de transférer artificiellement leurs bénéfices hors du pays où elle tire un revenu grâce au prix de transfert, le tribunal a mais sera-t-il de Paris ainsi jugé en juillet dernier que Google n'avait pas d'établissement stable en France et n'avait donc pas à subir de redressement fiscal, l'heure est venue en Europe de taxer les GAFA régulièrement accusée de faire de l'optimisation fiscale grâce à des montages financiers qui minimisent leur impôt, ils peuvent transférer leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, on y rémunérant des actifs incorporels et en profitant de conventions fiscales, la commissaire européenne à la Concurrence a récemment préconisé de fiscaliser Sega, derrière le dynamisme de ses gaffes à se cache une révolution qui peut provoquer de sérieux dommages collatéraux, prenons l'exemple d'Amazone qui a chiffre d'affaires égal emploi 5 fois moins de salariés plus Carrefour ou Casino, la progression de l'Amazone et fulgurante mais reste encore marginale dans l'alimentaire, on vient d'apprendre que ce géant américain cherche un cheval de Troie pour assurer sa conquête du marché français, Carrefour, Casino, Intermarché, Système U, aurait été approchés pour servir de tremplin cette firme pour l'instant, sans succès, mais on sait que ce développement est inéluctable, pas question de faire la fine bouche sur la nature des emplois créés ni de vouloir créer une impossible ligne Maginot pour protéger nos grandes enseignes nationales pour autant dérouler tapis rouge sans conditions à nouveaux prédateurs de la distribution, comme on l'a fait jusqu'à présent, pose question dans un autre domaine, ces firmes moyens gigantesques voilà autre question des droits sportifs TV jusqu'ici tenu par 2 chaînes de télévision payantes et les opérateurs télécoms aussi, Monsieur le secrétaire d'État au delà de la taxation gaffe que compte faire le gouvernement pour que ces entreprises soient soumises aux mêmes conditions que les nôtres, merci. La parole est à monsieur Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État en charge du numérique. Monsieur le président Monsieur, sénateur mesdames et sénatrice. Vous avez raison, la plateforme depuis quelques années on joué un rôle et joue un rôle de transformation notre économie majeure à telle point qui pose une question, une question essentielle c'est comment nos innovateur jouer avec plus d'égalité face à eux, ou avec, et quand je parle de nos innovateur, je parle de nos Start-Up, je parle aussi de nos PME, nos industriels de nos. Entreprises partout sur le territoire, je pense que la solution, elle tient en 3 piliers en 3 points, il y a le 1er qui celui sur la fiscalité, celui que vous avez abordé fiscalité les citoyens qui ne la demande des citoyens et patrons des PME, il le constate tous les jours il y a une inégalité, c'est bizarre de payer à ces plateformes autant et de les voir elle payé si peu en échange de la solidarité nationale c'est ce soutien populaire de tous les peuples d'Europe qui a fait que nous avons pu, avec le président de la République avec Bruno Lemaire, lancer une initiative lancée l'initiative avec les autres pays et leur proposer d'aller plus vite que l'agent d'international porté au sein de l'OCDE, dans lequel nous restons un acteur mais dont les résultats prendre encore quelques années plus vite encore que l'agent d'un Européen, avec la directive accises qui prendra elle aussi quelques années non, nous avons proposé une solution par cette taxe d'égalisation qui doit porter et nous espérons une solution dans les prochains mois dans les, dans les 24 prochains mois, sur ce sujet, il faut qu'on arrive à créer des majorités, aujourd'hui on parle déjà de 19 pays qui nous soutiennent, on a dit que certains ne soutenait pas et pourtant il y a 2 jours, j'étais au Conseil télécoms européen et ces pays qu'on disait ne pas soutenir ont rappelé leur engagement à trouver une solution pour cette taxation, je crois que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies et c'est encore une fois grâce aux peuples d'Europe aux citoyens qui se sont mobilisés, que nous sommes prêts à avancer mais il y a 2 autres sujets qui sont essentiels : le 2ème, c'est celui sur la transparence et la loyauté, et c'est pourquoi avec Bruno Le Maire, nous avons signé en début, au début du mois d'octobre, les décrets de la loi pour une République numérique qui vont apporter à tous les citoyens, plus de transparence dans les résultats qui seront affichés par ces mêmes plateformes aujourd'hui mais, enfin, et c'est le 3ème pilier c'est une invitation que je vous fais nous ont passé hier l'après-midi ensemble, certains d'entre vous pour un débat assez long sur l'Intelligence artificielle, la question c'est celle de nos en concluant Dick de concurrence et même de notre cadre de pensée il y a celui-là, je vous invite à l'venir à venir partager à venir participer à cet échange, parce que nous sommes en ce moment dans un jeu de prisonniers ou ces plateformes toute charmante quels sont attire les prix attire les prisonniers citoyen et les enferme dans des systèmes qui aujourd'hui empêchent les entreprises alors je vous y invite à participer à cette réflexion, c'est ce 3ème pilier-là qui nous permettra de préparer l'avenir. La parole est maintenant président Vincent et blessé pour le groupe socialiste et républicain chacun respecte les 2 minutes, y compris par Internet, merci. Merci Monsieur le Président, en l'absence de notre collègue Samia Ghali retardé par 100 vols depuis Marseille je me contenterai de vous lire sa question. Monsieur le ministre, cher Gérard Collomb la violence à Marseille est devenue banale et s'ancre dans le quotidien des Marseillais la bête se nourrit, et cette fatalité la république ne l'arrête pas dans cette bataille entre la loi de la rue et la loi de la République, chaque ministre dans son domaine, a le pouvoir, mais aussi le devoir d'agir car la délinquance, elle ne se met pas au chômage pendant que nous réfléchissons, au contraire, elle gagne du terrain, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours du président de la République sur la sécurité intérieure, sur cette question, je veux croire à sa volonté et à sa détermination, mais je m'interroge sur les moyens mis en face, la police de sécurité du quotidien à Marseille oui bien sûr, mais seuls pour intervenir dans les quartiers, elle sera inefficace et surtout en danger aujourd'hui, je suis inquiète pour la 2ème ville de France pendant que la délinquance s'enracine la méthode de l'approche globale lancée en 2012 est au point mort alors qu'elle commençait à faire ses preuves, les moyens humains et matériels ont régressé, y compris dans les zones de sécurité prioritaire les véhicules en 270000 kilomètres au compteur 6 équipages de la BAC quadrillent une ville de 850000 habitants, la sécurité publique a perdu une centaine d'agents en 2017 et à l'a perdu aussi 2 compagnies de CRS sur 3, je vous le demande donc, Monsieur le Ministre, car je vous s'est attaché à Marseille, dans quelles mesures le gouvernement est-il prêt à aider notre ville et quels moyens est-il prêt à mettre en oeuvre car sans sécurité, il n'y a ni espoir ni liberté pleine et entière et donc pas de république. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour vous répondre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices Monsieur je salue Samia Ghali évidemment sa question. Tout à fait pertinente quand on connaît les problèmes de Marseille oui, il faut assurer la sécurité qui est, je crois, l'une des principales préoccupations de nos concitoyens. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a de grandes préoccupations, me semble-t-il, dans notre pays à la fois le problème de l'emploi et ensuite celui de la sécurité, je pense que nous devons assurer la sécurité de nos concitoyens et c'est, comme vous le savez, une des priorités du président de la République, c'est pour cela que nous créerons 10000 postes de sécurité à la fois en police, gendarmerie et en services de renseignement au cours des 5 prochaines années mais, chers collègues, lorsque l'on regarde l'évolution des chiffres, on s'aperçoit, peut-être parce qu'il y avait eu la crise économique qu'entre 2007 et 2012 le nombre d'emplois dans les forces de sécurité avaient baissé de 12500 il a commencé à remonter à partir de la période 2013, 2016 avec 6500 emplois, emplois nouveaux qui ont été crées, c'est un et en 2017, ce seront 2280 6 emplois qui seront créés, enfin nous en créerons comme je viens de le dire 10000 emplois nouveaux, on pourrait annoncer à Madame Samia Ghali qu'à partir des sorties d'école qui vont se faire d'ici la fin de l'année ce sont 40 nouveaux policiers supplémentaires qui vont être réaffectés à Marseille, nous allons commencer effectivement dans chaque ville à remettre un certain nombre de forces de l'ordre et je pense que dans 5 ans nous aurons peut assurer les conditions de la sécurité du quotidien. Merci. La parole est maintenant notre collègue Pierre Charon pour le groupe, les républicains. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, ma question s'arrête à monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, monsieur le Ministre, il y a urgence à Paris l'annonce par le CIO de la qualification de Paris pour les JO 2024 a été une bouffée d'air pur, je dis bien une bouffée d'air pur, car la fermeture des voies sur berge à aggraver la pollution ainsi l'Observatoire indépendant sur la fermeture des voies sur berge dompte Airparif a rendu ses conclusions sans appel : le dioxyde d'azote ont bien augmenté alors qu'il reculait depuis 10 ans, ce type de mesures révèlent que Paris n'est malheureusement pas prête pour ce grand rendez-vous sportif à cause de certaines mesures prises par Anne Hidalgo, notre capital devient une ville musée, pourtant les valeurs de l'olympisme, ce sont le mouvement et l'action et non pas ce qu'il faut s'ils lisent notre capital. La circulation devient un exploit sportif, la seule discipline olympique spécifiquement parisienne, sans parler des autres courses d'obstacles que subissent quotidiennement les Parisiens avec sur l'écologie punitive, la maire de Paris, pénalise les faibles, cela fait fuir les parisiens les plus modestes, la volonté d'interdire les véhicules diésel, puis à essence n'est fait que pour satisfaire quelques bobos indispensables à la majorité municipale. L'économie de Paris est en péril, sans une circulation efficace les Parisiens d'Alès ainsi les petits et moyens commerces devenus inaccessibles, nous sollicitons l'aide de l'État. Pour mettre fin à ces mesures d'asphyxie incompatible avec ses qualités de capital organisatrice des JO, monsieur le ministre d'État, nous avons besoin de vous, et du préfet de police

Oui, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le Sénateur, Charon, vous auriez posé cette question à l'ancien maire de Lyon, il aurait pu vous répondra, mais aujourd'hui le ministre de l'Intérieur est un peu, si je puis dire, démunies dans la mesure où une loi du dit du 28 février 2017 a conféré les principales compétences en matière de voirie à la mairie de Paris et donc le préfet de Paris peut aujourd'hui faire un certain nombre de remarques mais sauf sur les axes, on va dire stratégique, il est aujourd'hui démunis il peut donner un certain nombre de conseils, mais c'est aujourd'hui le maire de Paris et le Conseil de Paris qui décide dans la perspective des Jeux olympiques, nous avons demandé, j'ai écrit personnellement à Madame la maire de Paris d'avoir une réflexion globale sur l'ensemble de nos de l'agglomération parisienne, en effet, comme vous le savez, les jeux olympiques vont se dessiner à la fois sur Paris intra-muros, mais également sur la 1ère couronne et donc il convient que nous ayons une réflexion globale sur les circulations à l'intérieur de ce grand secteur si nous voulons réussir, les jeux olympiques 2024. Merci, la parole est maintenant notre collègue Michel Forissier, pour le groupe, les républicains. Merci Monsieur le Président, Madame et messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire, la transition ils écologique est un des objectifs qui vous incombe, Monsieur le Ministre, les agences de l'eau doivent répondre à des défis d'une pertinence capital pour l'avenir de l'humanité à savoir adapter les politiques du changement climatique atteindra 100 pourcent du du bon état des eaux en 2027 réussir la prise en main de la vie m'a pris par les collectivités élargir nos compétences à la biodiversité et accompagner le financement du renouvellement des réseaux et lutter contre les fuites, les arbitrages budgétaires du gouvernement sont en parfaite contradiction avec les objectifs fixés, en effet, la réduction des Budgets successifs de leur de 30 la baisse des effectifs, d'une part, l'augmentation de 25 à 50 millions pour le financement de la viande française pour la biodiversité et un nouveau prélèvement ainsi chiffre qui tué par l'Office national de la chasse et de la faune, d'autre part nous perd monteront plus d'atteindre les objectifs, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, venir sur ses arbitrages et redonner aux agences de l'eau, les moyens de remplir leur mission est d'atteindre leurs objectifs. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Forissier, depuis que j'ai j'ai pressé, responsabilité, j'ai rencontré à 2 reprises l'ensemble des présidents et des directeurs des agences de l'eau, ma conviction qui ne connaît pas de source, pour d'autres interlocuteurs, sans faire de mauvais jeu de mots, on va pas s'en priver et que leur gouvernance par bah ça a du sens et doit être préservée, les agences, et vous l'avez évoqué constitue un fantastique outil au service des politiques de l'eau, mais vous l'avez évoqué vous-même également de la biodiversité, une fois qu'on a dit ça, et nous sommes que des évolutions sont néanmoins nécessaires. D'abord, les agences doivent avoir un rôle pivot dans la politique de l'eau et la biodiversité et c'est bien dans cet esprit qu'elles vont financer désormais entièrement les opérateurs, la biodiversité, l'Agence française de la biodiversité, les parcs nationaux et vous l'avez dit l'ONCF parce que le lien est évident entre la gestion de l'eau et les écosystèmes, vous m'interrogez sur les moyens, ceux-ci sont quand même importants au titre du 11ème programme nous prévoyons quand même plus de 12,6 milliards d'euros sur 6 ans c'est exactement une somme qui est intermédiaire par rapport aux 2 programmes précédents 13,6 milliards pour le 10ème programme et 11,4 milliards pour le 9ème programme pour l'année 2018 le plafond des redevances qui pourront être versées aux agences de l'eau devait être, il a été remonté de 2,28 millions de milliards d'euros à la demande des députés en contrepartie de cette hausse du plafond qui était demandée par les agences on a reconduit le prélèvement sur leurs fonds de roulement 200 millions d'euros, ce qui est à rapprocher leur trésorerie abondante par ailleurs de 760 millions d'euros, voilà la situation est cependant variable suivant les bassins sachez en tout cas que je veillerai à permettent à chacune de ses exigences d'exercer pleinement ses missions dans le cadre de ce 11ème, programme. Monsieur le ministre, je suis profondément déçu par votre réponse et puisqu'on en est aux yeux du monde, je vais vous dire monsieur le ministre, même si pour l'instant en France, on ne manque pas d'eau, je crains qu'à force d'avaler des couleuvres, vous prenez le risque de manquer d'air. Pour moi, vous savez, l'amendement qui a été présenté par le gouvernement au débat de l'Assemblée nationale est un leurre, parce qu'il prend et apporte un prélèvement supplémentaire au profit Direct de l'État 200 millions d'euros pour 2018, alors on donne un peu d'air maintenant et on le reprend après pour nous, Monsieur le Ministre, l'eau est source de vie, élément indispensable pour l'existence de l'homme sur la Terre, elle ne doit pas être considéré comme une base de fiscalité servant de facteur d'équilibre pour le budget de l'État, cette conception est un retour au Moyen-Age, où était prélever l'impôt sur le sel, symbole de leurs cadres, donc on a la fiscalité, l'eau est au contraire un bien commun qui doit être préservé comme Patrimoine essentiel pour l'humanité, merci. La parole est maintenant à notre collègue Annie Delmont police pour le groupe, les républicains, vous avez la parole, ma chère collègue. Merci monsieur le président, mes très chers collègues, ma question s'adresse à Madame Annie diffuse un ministre la c'est la des solidarités, de la santé, madame la ministre, le 13 octobre dernier, votre gouvernement a présenté son plan de renforcement de l'accès territoriale aux soins, ce qui a donné l'occasion à Monsieur le 1er ministre de déclarer que chaque citoyen d'avoir accès à une médecine de qualité, quel que soit l'endroit où il vit, de trop nombreux territoires où la densité médicale est inférieur de 30 pourcent à à la moyenne nationale souffre d'inégalités d'accès à la santé, la Seine-Saint-Denis se trouvent même dans une situation critique ce département manque cruellement de médecins et 45 pourcent d'entre eux sont âgés de plus de 60 ans, cette situation est la même dans de nombreux départements ruraux, le projet de modification de zonage ambulatoire pour l'aide à l'installation des médecins récemment présenté, ne fait qu'aggraver notre inquiétude : les nouveaux critères d'accessibilité ne rendent pas compte de la situation réelle des territoires par exemple des communes aisées de l'ouest parisien sont favorisés, alors que les territoires fragilisés du Nord-Est francilien ne sont pas considérées comme des zones prioritaires, vous n'avez pas les médecins de secteur 2 ce qu'il faut aux autres résultat dans les zones en difficulté quelque qu'elle soit rurales ou urbaines, il y a souvent que les médecins libéraux en secteur 1 qui exerce ce sont eux qui incarne la médecine de proximité, madame la ministre ma question est la suivante est-ce que la lutte contre l'inégalité d'accès aux soins de proximité dont souffrent tant la Seine-Saint-Denis fait réellement partie de vos priorités, ou bien allez-vous se laisser mettre en place une médecine à 2 vitesses, les plus démunis seront laissés-pour-compte. Pour vous répondent : la parole au secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je voudrais de nouveau excusé Madame Buzyn, qui est toujours au banc à l'Assemblée nationale pour défendre le PLFSS et je voudrais, puisque les ministres n'ont pas le droit de réplique rappeler que sur la question précédente, penser qu'il y a des solutions informatiques à tout aurait pu nous éclairer, quand on a mis en place dans ce pays, un logiciel qui s'appelle Louvois en 2011 et en 2021 on terminera en sortira enfin de cette difficulté, permettez-moi, plus globalement, de penser que c'est justement non pas des solutions informatiques qu'il nous faut inventer sur des sujets aussi essentiels que la présence médicale partout en France, que ce soit dans la ruralité ou dans n'importe quel quartier de votre département d'Île-de-France, il faut trouver des solutions appliquées au terrain, il faut faire confiance à l'Intelligence collective du territoire il faut pas penser à la coercition, certains imaginent qu'on pourrait imposer des présences imposer des installations médicales pour les jeunes médecins, ce serait faire fuir l'installation mettent de médecins et l'engagement dans la profession de médecin mal inverse : nous voulons chercher au plus près du terrain, toutes les solutions à travers un plan ambitieux qu'a présenté le 1er ministre et Madame la Ministre de la Santé qui se construit autour de la volonté de renforcer les coopérations, notamment en doublant le nombre de maisons de la santé, elles ont fait leurs preuves, elles marchent, elle fonctionne, il faut aller plus loin, il faut pas penser que c'est la solution à tout, mais c'est un élément important et dans les quartiers comme dans la ruralité, il faut renforcer ce dispositif, il faut aussi développer les capacités d'intervention sur l'ensemble de la chaîne médicale et le dispositif azalée qui permet aux infirmières infirmières de prendre en charge des maladies chroniques, sous l'autorité d'un médecin doit permettre aussi d'alléger sur sur certaines fonctions, la charge de travail des médecins, il faut aussi développer les pratiques avancées qui sont essentiels et qui permettront à des professionnels d'exercer au-delà de leur spécialité initiale dans le même esprit, nous voulons encourager l'innovation et notamment la télémédecine par la possibilité de rémunérer le médecin qui fait un acte à travers la télémédecine et nous voulons plus d'incitation en simplifiant la vie administrative des médecins pour qu'il passe l'essentiel de la réactivité, non pas à faire de la paperasse, mais à accompagner les femmes et les hommes dans vos quartiers comme dans l'ensemble rurales pour faire en sorte qu'on puisse améliorer et garantir un vrai accès aux soins. Merci monsieur le ministre, j'espère donc que vous ne maintiendrait pas les critères que j'ai pointé du doigt et qui conduisent à une situation inégalitaire j'en appellerai toujours à l'application du principe d'équité qui seule peut endiguer l'inégalité d'accès aux soins dans les territoires fragilisés un exemple supplémentaire le démantèlement programmé de l'hôpital Jean Verdier de Bondy pour lequel tous les élus de Seine-Saint-Denis, toutes tendances confondues, sont en alerte et seront vigilants pour que l'accès aux coureurs soit garantie sur le territoire, la défense de la Sambre, n'a pas de couleur politique, elle doit garder garder des solutions technocratiques Mes chers collègues, les prochaines questions d'actuel, et auront lieu le 31 octobre à 16 heures 45 je remercie Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les ministres, de leur présence les suspende la séance, elle sera reprise à 16 heures 30 pour un un débat. Sur le logement social. Sûr qu'elle territoire comment et pour qui, demain, la séance est suspendue.

Merci, mes chers collègues, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat logement social sur quel territoire comment, pour qui demain. C'est une demande du groupe de l'Union centriste. nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur du débat disposera d'un temps de parole de 10 minutes, y compris la réplique. Puis le gouvernement répondra pour une durée équivalente. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat, il s'agit de monsieur Daniel Dubois pour le groupe de l'Union centriste pour 10 minutes. Monsieur

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis plusieurs semaines, le mouvement HLM auquel se sont associés les professionnels du bâtiment et les associations de locataires, tire la sonnette d'alarme la demande qui est faite aux bailleurs sociaux de compenser la baisse de l'APL par une baisse de leurs loyers va les priver un 1000000000 7 d'euros de recettes. Dès 2018. Le pronostic vital d'environ 200 organismes sera engagée. D'ici 5 ans. C'est l'intégralité des bailleurs sociaux qui sera en grande à cela s'ajoute. Dans le projet de loi de finance l'augmentation de 100 millions des cotisations Hoffmann, ainsi que le gel des loyers en 2018 pour un un manque à gagner d'environ 150 millions d'euros. Ce sont donc. Mais, chers collègues, 2 milliards d'euros de ressources qui vont manquer au logement social.

Y compris dans le secteur privé. Puisqu'une partie des opérations sont mixtes et vendu en VF a. Nous connaîtrons également. Un ralentissement des réhabilitation énergétique, ainsi qu'une réduction drastique des crédits d'entretien. Et le gouvernement, Monsieur le Ministre, hausse parlé d'un choc de l'homme. Je suis désolé de vous dire. Que c'est plutôt un choc dans le mur alors que vous êtes en train de nous préparer. Le gouvernement s'est enfermé dans une logique purement comptable. Qui pêche par son uniformité alors même que les situations des bailleurs sur nos territoires sont diverses. Une logique au demeurant totalement injuste. Puisqu'elles ponctionnent les 9 milliards d'APL versées dans le secteur HLM sans s'interroger sur les 9 autres milliards d'euros versés cette fois-ci dans le secteur privé. Il semble. Que de telles considérations non pas encombrer le gouvernement. Il a besoin d'un 1000000000 et demi pour équilibrer son budget et la mesure sur l'APL peut lui rapporter ne rapporter près de 2. Permettez-moi d'indiquer. Que ce n'est pas l'amélioration des conditions d'emprunt. L'augmentation inapplicable des surloyers ou encore la vente de logements à des locataires impécunieux qui permettront de compenser une telle perte. Alors je devine évidemment Monsieur le Ministre, les arguments du gouvernement, le président de la République a lui-même déclaré, et je reprends ses mots qu'il a 2 problèmes avec les HLM premièrement, le trop grand nombre d'opérateurs qu'il estime à 800, notons au passage que l'USH ne recense que 519 organismes dans le domaine du locatif social, deuxièmement la mauvaise circulation du capital avec des organismes qui aurait des trésors sans construire dès et chers collègues, la volonté du gouvernement apparaît clairement phase 1 il appauvrit les bailleurs efface 2 il livre les plus fragiles à l'appétit les plus solides, voilà la stratégie pour le logement, demain, si nous n'y prenons pas garde, ainsi on réduit drastiquement le nombre d'organismes ainsi laissé les capitaux circulent alors circulez, circulez, il y a plus rien à voir. Monsieur le Ministre votre moralement, a-t-il bien conscience des conséquences qu'aura sa politique est-il conscient de son impact sur l'emploi. Les HLM génèrent 17 milliards de travaux par an. Mobilise l'équivalent de 170000 emplois non délocalisables dans le secteur du bâtiment et souvent d'ailleurs de manière contracyclique, le gouvernement Monsieur le ministre est-il conscient. De son impact sur la fiscalité, chaque année, les organismes HLM acquitte un 1000000000 d'euros de TVA. Le gouvernement est-il conscient, Monsieur le Ministre que faute de bailleur, l'article 55 de la loi SRU va devenir inopérant le gouvernement Monsieur le ministre est-il conscient du risque encouru par les collectivités territoriales en cas de mobilisation des garanties d'emprunt. Le gouvernement est-il conscient, Monsieur le Ministre, que les organismes ne pourront plus s'engager dans la rénovation urbaine, alors même qu'ils avaient financé 45 pourcent du du PNR hein, soit 3 milliards d'euros sur leurs fonds propres. Le gouvernement est-il conscient, monsieur le ministre, enfin. De la fracture sociale et territoriale, qu'il va exacerber en créant des organismes de Taiji, grand qui siphonne rompt les loyers des territoires périphériques pour construire en zone tendue, monsieur le Ministre. Baisser drastiquement l'APL revient à déstructurer tout le secteur du logement social, sans que nous en discutions. Sans une bribe de débat et sans vision d'ensemble, je crains pour tout vous dire, un à croyable rendez-vous manqué. Permettez-moi d'identifier un problème de méthode comme cela que nous réformons dans notre pays. Sans concertation. En marche forcée avec des objectifs budgétaires mais sans stratégie pour le secteur. Permettez-moi ensuite. Monsieur le ministre, de pointer une vraie méconnaissance du monde HLM. Face aux millions de chômeurs, de ports de mal-logés, face aux défis de l'aménagement équilibré de notre territoire, le logement aidés est au coeur de notre pacte social. Il mérite un débat plus large qu'un débat budgétaire. S'il doit être réformé, cela ne peut pas être au détour d'un article du projet de loi de finances. Profitons d'être à la croisée des chemins pour nous poser des questions fondamentales. à quoi doit servir le logement social. Alors uniquement les plus défavorisés ou à organiser la mixité sociale, il s'agit là d'un véritable débat de société, comment doit-il fonctionner, quel est le rôle de l'État, après s'être désengagé de la la la construction doit-il ne plus contribuer à la solvabilité des ménages j'aimerais, monsieur le ministre, avancé quelques propositions, ne soyons pas uniquement fixées sur les économies à réaliser, certes, le logement social doit pouvoir être plus efficient, nous ne mettons pas cela en cause, mais il peut aussi bénéficier ou générer de nouvelles recettes réfléchissons à la manière dont nous pouvons drainer de l'argent privé vers le logement social par le biais de dispositifs de 10 fiscalisation par exemple, la Fédération des eaux propos responsable par une hausse conséquente de la TVA sur la construction de logements neufs, réfléchissons à la mise en oeuvre de 2 stratégies distinctes en fonction des territoires, l'une axée sur la production massive de logements en zones, l'autre sur l'équilibre du territoire et le renouvellement des populations zones périphériques ou rurales en élargissant les compétences des organismes au jeu autour d'objectifs partagés la revitalisation des centres bourgs, les services à la population l'ingénierie auprès des collectivités, à optimiser le traitement de la demande de logement par le biais, par exemple de plateforme nationale dont l'objectif serait la garantie d'une attribution suite à une mutation professionnelle réfléchissons aussi ont bâti depuis la loi de 2005 sur l'accessibilité, par exemple, on assiste à une des densification des constructions, alors même que le prix du foncier est un enjeu majeur, 2 tiers des nouveaux immeubles dépasse pas 3 niveaux, la plupart des logements sont accessibles, ce qui génère des surcoûts, pourrions-nous réfléchir à des immeubles avec une mobilité assurer quel qu'en soit la hauteur et à des logements vraiment évolutif, vous voyez, Monsieur le Ministre, ce débat peut être passionnant et des solutions sont envisageables, je vous propose donc dans l'immédiat et face à l'urgence budgétaire que vous puissiez vous engager à réécrire l'article 52 du projet de loi de finance en bonne Intelligence et en lien avec tous les partenaires, le Sénat s'honorerait de participer à untel exercice sachez par ailleurs qu'il est très sensible à la problématique du logement dont la réalité se vit tous les jours dans les territoires, il sera toujours disponible pour débattre et contribuer à une réforme globale en conclusion, Monsieur le Ministre, vous aurez compris mon message ne prenons pas le risque de déstabiliser durablement un secteur qui recouvre tendant je me socio-économique ne passons pas à côté d'une vraie réforme pour réaliser des gains relatifs si on considère l'effet de levier du logement dans notre pays, j'espère que vous n'entendrez et merci de votre attention. état monsieur Julien Denormandie ça. Ces Terres d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires pour une durée de 10 minutes environ. Monsieur le président, Mesdames sénatrices messieurs les les sénateurs, je vais essayer de répondre dès mon propos introductif à beaucoup des points que que vous avez évoqué, monsieur le sénateur du bois. La première chose et je le dis avec énormément de conviction et aussi de fermeté, le gouvernement ne cherche en rien à déstabiliser le secteur d'HLM rien. Et je le dis avec d'autant plus de fermeté, Pour toutes celles et ceux qui ont pu avoir des échanges avec ces organismes avec ces sociétés et savent que les discussions que nous ce que nous avons avec avec nous les avons depuis le 1er jour nous les avions d'ailleurs entamé bien avant le débat sur les affaires bien avant et nous les avons toujours eue avec un seul souci de se demander comment fait-on pour résorber résorber la situation actuelle où effectivement il n'y a pas suffisamment de logements sociaux en France, on a entendu tout et son contraire sur le sujet, on nous a d'abord pendant l'été, accusé une ou le gouvernement de vouloir revenir en arrière sur la loi SRU, on nous a ensuite dit que le gouvernement pour

à la fin, au bénéfice des locataires j'ai reviendrait donc oui Monsieur le sénateur, le pouvoir, le gouvernement est conscient de la nécessité de préserver le modèle du logement social, oui, Monsieur le Sénateur, le gouvernement est conscient de l'enjeu de la rénovation urbaine, et le gouvernement sait très bien que la rénovation urbaine, c'est pas financé uniquement par l'État, c'est pas financé uniquement par l'Union sociale habitat ou par la par Action logement c'est financé par les bailleurs eux-même qui, à la fois contribue au programme de l'ANRU mais surtout à chaque fois que l'enrhumé 1 euros financé par de la dette supplémentaire, les projets de rénovation urbaine. L'engagement de l'État sur la rénovation urbaine, on en reparlera pendant les les questions qui suivra nos propos introductif, l'engagement de l'État sait mettre un 1000000000 d'euros pour doubler, in fine, et le nouveau programme de de l'ANRU un 1000000000 d'euros, ce fameux 1000000000 d'euros, dont on entend parler depuis des années et qui n'avait jamais été budgétés, on le fait, puisque le projet de loi de finances inscrit déjà ses premiers crédits dessus, oui Monsieur le le sénateur, le gouvernement est aussi conscient que le système actuel, il n'est pas optimal n'est pas suffisamment efficients et que des choses peuvent être faites, oui, Monsieur le Sénateur, le gouvernement est conscient que les différents offices des différentes sociétés non absolument pas les mêmes caractéristiques non absolument pas les mêmes solidité de bilan non absolument pas les mêmes capacités d'emprunt non absolument pas les mêmes niveaux de ressources et même plus, non, absolument pas la même attention vis-à-vis d'un public social ou d'un public qui a été très fortement quand vous prenez le taux de personnes aux APL il diffère de manière significatif entre Office ou entre sociétés significative, vous pouvez avoir des offices avec 15 pourcent de de personnes aux appels et d'autres avec 75 ou 80 d'ailleurs souvent ceux qui ont le plus de personnes aux appels sont ceux qui sont souvent dans des situations financières plus difficiles et souvent dans des territoires qui ont trop souvent été oubliées donc si le gouvernement en a pleinement conscience et le gouvernement dans tout ce qui fait prendre cela en considération. Eh oui, enfin Monsieur le le sénateur, le gouvernement est attaché une méthode, une méthode de discussion, une méthode de concertation, je l'évoquais tout à l'heure, comment Madame la sénatrice, Estrosi, ça, ça ne m'interroger. Au 1er jour lors de nommer notre nomination avec Jacques Mézard, on a rencontré les bailleurs sociaux, j'étais encore avec, hier soir, j'étais encore avec ce matin, je les vois absolument tous les jours ou tous les 2 jours, dans ce souci de concertation et de et de discussions, pourquoi, aujourd'hui, la situation peut-être amélioré je vous prendre quelques exemples, et je vais vous parler vraiment en toute franchise et en toute transparence. On a évoqué avec l'ensemble des bailleurs sociaux un certain nombre de pistes de travail, la première pistes de travail. C'est de de voir comment vous pouvez améliorer le financement des opérations de logements sociaux, je prends 2 exemples, aujourd'hui, on le sait bien, un logement social c'est financé uniquement sur un apport de capital et de la tête par les bailleurs et cette dette est apportée par l'État, plus précisément, la Caisse des dépôts, avec une contre-garantie, les collectivités locales, qui est un point essentiel est très important, il s'avère que tous ces outils-là en tout cas dans son son aspect de financement, il est dans il est dans les mains de l'État et de et de la Caisse des dépôts, notamment, et donc on a entrepris un travail parce que ça les bailleurs sociaux oublient souvent de vous le dire mais demandez leur, on leur a communiqué à chacun, à chacun, l'État est entré avec avec avec un souci, c'est de savoir comment on pouvait améliorer ses opérations de financement des exemples, là aussi, très précis, les bailleurs sociaux nous disent : nous on veut des prêts de votre bilan, alors je vais pas rentrer dans la technicité mais ça permet d'avoir plus de capital et donc c'est un élément très bénéfique, passé 2 milliards pour leur proposer, ils nous disent aujourd'hui, on ne peut s'endetter que avec des prêts à taux variable pour les financiers que vous êtes ces prêts à taux variables, ça veut dire que chaque année, vous ne savez pas comment vous, vous pourrez pas quels seront le les sommes que vous devrez verser, hé bien on leur propose pour la première fois des prêts à taux fixe, avec des remboursements qu'on appelle in fine ça veut dire que le remboursement n'intervient qu'à la fin, c'est un impact Direct sur leur trésorerie nous disent : il faut améliorer notre capacité à rénover énergétique, c'est 3 milliards d'euros qu'on leur propose 3 milliards d'euros, ils nous disent aussi dans, dans certains cas, il faut qu'on puisse avoir des allongements de près et que d'ailleurs si vous nous proposez d'annoncer ce prêt parce qu'on le fait à hauteur de 30 milliards d'euros, 30 milliards, ça n'a de sens que si le coût supplémentaire d'un allongement qui soient pris en charge par l'État et par la Caisse des dépôts, alors on leur a répondu OK, on est prêt à à en discuter pour que ce sur sur à terme parce que bénéficie, mois par mois, ce sur quoi, à terme, sera pris en charge par l'État et la Caisse des dépôts,

qui est inflationniste possible et qui n'est pas pérenne, alors on peut, on peut dire ce qu'on veut, on peut se dire on continue à vivre comme ça, avec le système des appels, c'est pas pérenne, il y a une erreur fondamentale qui a été faite à la fin des années 70 qui a été de se dire : on passe d'une aide à la construction à une aide au logement, elle, était sûrement juste à des pop, mais la conjoncture économique qui s'en est suivie a montré qu'en faisant ça, en fait on a cessé d'accroître les aides personnelles au logement et donc ce qu'on dit aux bailleurs sociaux, c'est tout ce gain supplémentaire que vous avez, il faut qu'en revanche on puisse ensemble. En faire à la fin, profiter le mécanisme tout entier désagréable et donc de participer à la diminution de ces charges qui aujourd'hui représentent 18 milliards d'euros, 18 milliards d'euros, c'est la moitié du budget de l'Éducation nationale

au 1er jour avec l'ensemble des organismes HLM notamment leurs représentants, on aurait dit est-ce que on peut ensemble travailler sur cette accession sociale, c'est-à-dire permettre à certains de pouvoir acquérir leur logement, mais pourquoi on radie ça

C'est 4 millions et demi de logements qui sont valorisés à 0 dans les comptes de tous les offices et toutes les sociétés, pourquoi, parce qu'il est réputé, que vous ne pouvez pas les vendre certains économistes disent que la valeur de tout cela, c'est 230 milliards certains,

le plus proche de logements intermédiaires ou du logement privé, mais c'est à peu près 20 pourcent donc donc sur les 4 millions et demi ça peu près de 900000 logements à l'intérieur de ces logements, il y en a pas tous, mais il y en a qui souhaitent pouvoir acquérir leur logement, c'est encore d'autres difficultés, qu'il faut régler des difficultés copropriété par exemple ces difficultés de copropriété, il faut apporter des solutions, imaginons qu'aujourd'hui vous avez donc 4 millions et demi de ménages à peu près grosso-modo 900000 ménages qui sont dans ce qu'on appelle ces logements de PLS. Chaque année, on va un peu près 8000 logements 8000 simplement sur lequel, si demain on passait à 20000 logements, imaginons, imaginons que 20000 logements ça représente à peu près 100000 euros, un logement, ça fait 2 milliards d'euros, le revenu annuel donc je parle de 20000 logements sur 4 millions 5, le revenu annuel. Total des bailleurs sociaux, c'est-à-dire les loyers qui perçoivent, c'est un peu plus de 20 milliards ce 2 milliards c'est 10 pourcent Et ça c'est un vrai sujet de travail qu'on a une vraie piste d'un 1000000000 d'améliorations qu'on a avec eux, parce qu'à la fin, ça fait quoi ça permet de rentabiliser une opération beaucoup plus fortement et de diminuer les loyers pour les locataires pour les bénéficiaires et je parle bien là d'accession sociale, je parle pas du tout de vente à des institutionnels ou autres, je parle vraiment d'accession sociale et donc ça ce volet là c'est une 2ème piste de travail qu'on a avec eux et sur lequel beaucoup sont tout à fait enclin à travailler en ce sens et d'ailleurs, dans le projet de loi et ce sera un sujet sur lequel il faudra qu'on qu'on qu'on travaille avec vous dans le projet de loi de logement on apportera les modifications pour faciliter cette accession sociale 3ème sujet je, je, j'essaie d'être rapide 3ème sujet. ça concerne le regroupement que vous avez évoqué, monsieur le sénateur du bois ce regroupement, il est aujourd'hui appelé de ses voeux par les organismes et des sociétés HLM, on a beaucoup discuté avec eux, il y a appelé de leurs voeux par eux-mêmes, pourquoi, parce que c'est plus de possibilité aussi d'accueillir des gens avec plus de difficultés financières, quand j'ai évoqué tout à l'heure, ces disparités d'un bailleur social à un autre, mais il faut aussi rassembler alors ça dépend ce qu'on a ce qu'on appelle rassembler beaucoup se sont organisés en GIE, par exemple, d'autres se sont vraiment solidifier dans des groupes en tout cas, il faut rassembler pour pouvoir accueillir aussi des publics plus sensible quand justement certains n'ont pas la capacité de de les accueillir, mais c'est aussi plus de capacité financière à la fin pour pouvoir mieux construire et enfin dernier point sur ce volet du logement social, monsieur le sénateur que que vous évoquiez une fois qu'on a parlé du financement, une fois qu'on a parlé du du de la vente, une fois qu'on a parlé du regroupement, il y a effectivement cet article 52 de du projet de loi de finances, l'article 52 du projet de loi de finances, c'est l'article sur lequel nous négocions aujourd'hui avec l'ensemble des bailleurs sociaux, comme comme vous l'indiquez est vraiment en toute transparence, en toute franchise, on ne on en discute, absolument tous les jours, les bailleurs sociaux nous ont dit au début, ce que vous nous avez proposé notamment les améliorations de financement, ça ne convient pas, on a continué à travailler, on leur a, on les a revus, on leur a écrit, et c'est le 1er ministre lui-même qui l'a fait et, aujourd'hui, de même il voit des avancées significatives sur ce package financier, ça ne leur convient toujours pas je vais pas me cacher derrière une contre-vérité, ça ne leur convient toujours pas, je pense que la presse, les campagnes de pub qui finance mais on a aujourd'hui devrait pistes de travail avec eux, je veux donner des exemples comprend revenir dans les questions, il trouve que l'article 52 qui repose que sur une baisse de loyer et peut-être trop rapide, vous l'avez évoqué monsieur de sénateur, il nous demande si on peut évoluer, par exemple, sur des sujets tels que la taxation comme la TVA, parce que pour eux, c'est plus de souplesse, plus de de simplicité pour monter en puissance, on est en train de travailler avec le dessus si ça peut permettre à terme de baisser effectivement la dépense des APL, mais de le faire de manière plus progressif en travaillant sur la TVA, donc ça on on on a rediscuté encore hier soir avec encore ce matin, c'est une piste de travail sur lequel on avancera, je reviendrai dans les questions, je veux pas être plus long parce que le temps qui m'est imparti est révolu, mais je voulais juste également insister sur 3 derniers points, vous avez évoqué, monsieur le sénateur, beaucoup de pistes, en appelant le gouvernement à pouvoir y répondre positivement, parmi toutes ces pistes, il y en a beaucoup qu'on fait déjà et sur lequel nous sommes totalement aligné, j'ai noté, notamment la TVA, je viens d'en parler, j'ai noté la rénovation du centre bourg notre conviction avec Jacques Mézard centre bourg notamment la rénovation des centres villes, de villes moyennes, a été l'un des terribles des dernières années et donc dans toutes les négociations que nous avons fait, nous sommes en train de de lancer un plan logement de rénovation qui est déjà en construction depuis maintenant 2 mois et nous avons notamment obtenu d'Action Logement qui puisse financer à hauteur de 1 1000000000 5 sur 5 ans, la rénovation des centres bourgs de villes moyennes, parce qu'il faut en faire un axe fort de la politique du logement, vous avez évoqué également monsieur le sénateur, les systèmes de plateformes, il y a aujourd'hui une plateforme d'attribution qui s'appelle des plateformes je d'accord avec vous, il faut voir comment on peut améliorer le le système, vous avez en enfant enfin, ils

parce que le système du logement dans le secteur privé, notamment il y a un truc qui est aberrant, c'est que les intérêts des uns et des autres, ils ne sont pas dignes dans la vie, quand les intérêts sont pas quand les vents sont contraires à la Marie hé ben vous avancez pas vous fait du surplace et typiquement, c'est pour ça qu'on va faire un abattement fiscal massif avec si moi, en tant que citoyen, cherchant un logement, j'ai besoin d'terrain mais certains d'entre vous, en tant que propriétaire vous n'avait pas intérêt invente parce que si vous attendez 22 ans avant de vendre à ce point-là, vous paierez pas de d'impôt sur la plus-Value immobilière le truc qui va pas marcher et donc ce qu'on dit c'est tout

alors je pense qu'on fait la même chose avec les entreprises et c'est également un des axes de de travail que nous avons dans le cadre de la conférence nationale des territoires, enfin vous évoquiez les logements évolutifs logement et évolutif notamment beaucoup travaillé avec notamment l'APF, l'Association des paralysés de France et nous sommes avec eux, tomber sur un schéma global de ce que doit être un logement évolutif, nous l'avons définie avec eux sur ce dernier point, je pense qu'il y a ce sujet mais qu'il faut pas non plus se tromper d'objectif, le vrai sujet de l'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap, c'est pas que les logements neufs, c'est avant tout les logements existants, et notamment les logements publics quand vous voyez que notre ministère aujourd'hui n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap, je suis mal placé pour donner des consignes aux uns et aux autres en disant soient enfin prises alors que mon ministère lui-même, n'est toujours pas accessible, je vous remercie. je serais un petit peu plus directive sur le temps de réponse, c'est le temps d'expression. Donc le 1er orateur c'est Monsieur Abdallah Hassani pour 2 minutes. Ce monsieur le président, monsieur le ministre, je suis un peu inquiet, les propos que j'ai entendu ici. Je me rends compte que sur le plan national, il y a un déficit de logements sociaux. Que dire de l'Outre-mer. Et particulièrement de Mayotte, vous savez que le parc de logements sociaux à Mayotte, et de 300 seulement 300 pour une une population de pratiquement 300000 habitants avec. 10000 naissances. Laurent, vous imaginez le retard qu'on a à Mayotte. Par contre, il y a des efforts qui ont été faites quand même. Les conditions techniques. Pour produire durablement son temps présent réunis. Des projets et des opérateurs sont prêts, l'établissement public foncier et d'aménagement qui n'existait pas, a été mis en place en juin dernier pour améliorer, pour améliorer l'acquisition du foncier et le réseau des dessertes. De freins au développement des constructions à Mayotte. Mais le financement ne suit pas Monsieur le ministre. implicitement foncier n'de doté, autres que de 3 millions d'euros seulement par an pour 5 ans. Et ce montant et épreu levé sur la Ligue budgétaire unique déjà très insuffisantes. à laquelle le ministre des Outre-mer : contribuer à l'amélioration de l'habitat. à Mayotte, elle ne recouvre pas les besoins de la seule intercommunalité Mamoudzou Déndéni. Soumise à la loi SRU. à l'obligation de produire 888 logements locatifs sociaux. En 2019, c'est pourquoi je vous pose la question. Comment le gouvernement prendra toute sa part au développement du logement social à Mayotte. Merci. Si le président, Monsieur le Sénateur, effectivement aujourd'hui le la situation que j'évoquais sur le logement social, site si elle est pardon compliqué en métropole, elle est souvent encore encore plus et voir bien plus compliqué, dans un certain nombre de territoires tous trentenaires, je prends des exemples très très concrets, on sait que par exemple il y a eu des sujets intenses, de longues discussions sur les sites de avec son actionnariat avec la présence d'un certain nombre d'actionnaires, on savait plus qui faisait quoi, alors qu'il fallait aller de l'avant et développer trop souvent on a eu des débats qui qui étaient des débats de de structures institutionnelles et pas des débats qui visait à délivrer, comme vous l'avez rappelé monsieur le sénateur, effectivement, grâce au travail conjoint, on a pu mettre en place, notamment l'établissement, dit cette femme aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'il est suffisamment doté ou pas, d'autant plus que son financement est assuré par des lignes budget directement du ministère des Outre-Mer ce qu'on appelle la ligne LB et qui en limite son son financement alors 2 éléments de réponse le 1er c'est qu'il y a tout un travail qui est en cours pour essayer de voir comment on peut évaluer et les répartir spécifiquement les besoins d'un territoire à l'autre pour voir là où il faut mettre l'accent quant à quant au déploiement de cette ligne budgétaire, ce travail est en cours avec le ministère des Outre-mer le de le 2ème, le 2ème élément, le 2ème élément, c'est que, au-delà des capacités de financement de de la femme et de tous les débats publicitaire qu'il y aura notamment dans les lois de finances, je pense qu'il y a un acteur, mais si vous l'avez évoqué mi-mai succinctement, c'est le travail de l'ANRU et notamment le travail de l'ANRU dans le cas du NPA est rue aujourd'hui sur Mayotte, ces 3 projets qui sont financées la vraie question qu'il faut se poser parce que c'est là où vous voulez accroître significativement et massivement à une construction il faut vous passiez par des opérateurs tels que l'ANRU et pas uniquement par des lignes budgétaires, donc la question c'est : comment on va encore plus loin dans le déploiement grâce à un opérateur comme l'ANRU dans le cas du PNR formation. La parole est à la présidente, et il y a un assassinat pour 2 minutes. Merci monsieur le président, monsieur Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier le groupe Union centriste pour le choix du sujet de ce débat à l'heure où les contours du projet de loi sur le logement ont été dévoilés et donc à l'évidence, ce projet de loi va encore à aggraver la situation des locataires en précarisant lors droit avec la perte du maintien dans les lieux et les voies de l'extension de l'application du surloyer dans le même mouvement, votre gouvernement, monsieur le ministre a annoncé une baisse brutale des subventions aux collectivités qui sont pourtant des acteurs essentiels du logement social, une baisse brutale des aides à la Pierre, ainsi qu'une ponction indue sur les offices HLM qui devront prendre en charge les appels, le gel des crédits du budget de la politique de la ville, pèse également fortement sur la politique du logement à cela, ajoutons le gel du taux du Livret A, alors que c'était pas une finance la construction, c'est une attaque sans précédent contre le modèle social du logement public ces mesures rendent impossible la réalisation des missions d'intérêt général des bailleurs sociaux et concrétise le désengagement de l'État, dois je vous rappeler quelques chiffres quand même alarmant alarmant du mal-logement dans notre pays 4 millions de nos concitoyens sont mal logés, compte 12 millions sont en situation de fragilité 79 pourcent des des Franciliens sont éligibles au logement social, quand 600000 effectue une demande chaque année, défendre le logement social, c'est une exigence or la seule option encouragée par le gouvernement, c'est la vente par les bailleurs de leur Patrimoine pour être en mesure de continuer à financer la construction est-ce vraiment sérieux lorsqu'on connaît l'ampleur du nombre de demandeurs, diminuer le nombre de logements sociaux Est-ce là votre réponse à la crise du logement, comment dans de telles conditions, garantir le droit au logement pour tous. Madame la sénatrice, je suis désolé de vous dire, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de contre-vérité dans ce que vous avez dit dans votre question, très sincèrement, le maintien dans les lieux, on a toujours dit, je le redis, un instant ce qu'on ce qu'on propose c'est d'introduire de la de la mobilité en disant tous les 6 ans tous les 6 ans on proposé sa vie, il y a une une caisse d'attribution des logements, on dit que cette caisse d'attribution des logements, elle proposera tous les 6 ans, je, je, je, utilise le mot proposé aucune obligation, elle proposera locataires, s'ils le souhaitent, non ça ne se fait absolument pas ben je vous assure que ça ne se non, je vous assure que ça ne se fait pas et tous les 6 ans, elle le propre, ils pourront accepter ou pas, donc le maintien dans les lieux, il était évidemment fait vous dites que, est ce qu'il faut la solution, c'est diminuer le nombre de de demandeurs de logements sociaux vous expliquer, il y a absolument 2 minutes que justement on avait décidé de ne jamais utiliser cette aberration que serait de diminuer les loyers d'éligibilité le montant de revenus d'éligibilité au système social jamais donc ne concluait pas avec une telle affirmation, alors que je viens de vous expliquer que ça n'était pas le cas, enfin ville, la politique de la ville, l'ensemble des crédits de la politique de la ville, on les maintient sur la durée du quinquennat on a annoncé il y a quelques semaines sur le logement d'abord parce que là on parle que des bailleurs sociaux et vous évoquez les mal-logés

intermédiation locative 10000 pensions de famille, prenez les propos, y compris des associations de logements, d'abord du droit au logement qu'on voit, on a encore passé la matinée avec eux, il salue le programme de logements, d'abord porté par ce gouvernement, il le salue donc on peut pas dire que le gouvernement ne fait rien au bénéfice des mal-logés, bien au contraire, on a je crois un programme très ambitieux sur ce sujet je crois. Si Monsieur le Ministre. La parole est à la présidente Valérie Létard.

qui peut être une véritable bombe à retardement pour des raisons budgétaires que l'on peut comprendre l'État de maîtriser sa dépense publique, mais avec des effets collatéraux massifs sur les risques de fracture territoriale et sociale que peut générer une situation comme celle-ci, je vais pas rappeler tous les chiffres, vous l'avez fait tous les uns et les autres, mon collègue Daniel Dubois rassembler tous les sujets, tous les risques qui étaient ceux-là, moi je voulais vous parler particulièrement de l'ANRU

il va falloir ensuite, contribuer, accompagner le FNAP au niveau du USH cela va forcément diminuer les fonds propres des désirs des organismes bailleurs qui vont devoir faire des choix rénover thermiquement leur logement, construire un petit peu de logements nouveaux, allez sur l'ANRU, on voit bien qu'ils pourront pas tout faire, vous nous dites : ventes de Patrimoine, on a créé des sites en rue pour gérer les copropriétés dégradées liées à la vente de Patrimoine, donc oui il faut faire quelque chose, Monsieur le Ministre, on en est convaincu mais profitez du travail parlementaire qui va être fait ici au Sénat, vous avez vu sur tous les bancs, tout le monde est convaincu qu'il faut avancer dans le bon sens monsieur Ministre mais sur l'ANRU si on veut pas que les 5 milliards annoncés dans le 1000000000 de l'État ne soit pas une chose que de l'affichage parce que les collectivités, elles vont peut garantir un emprunt parce qu'on va déjà les venir les chercher sur leur propre garantie aujourd'hui, elles vont devoir payer la CGT laisse aujourd'hui ne pourra pas assumer avec le peu d'argent qu'elle a et derrière les collectivités seront mobilisés à hauteur de 50 pourcent de de ce qu'il faudra faire quand on aura mis en croire les bailleurs, bref, tout ceci pour dire que maintenant il va falloir, monsieur le ministre, reconstruire un article 52 qui nous permettent, hé bien de trouver des solutions attend dehors de refonder une politique de logement et de la rénovation urbaine, en commençant par le commencement et non pas en rabotant le budget pour raboter le budget en mettant encore une fois en croire quelque chose qui doit s'améliorer, mais qui est indispensable pour que les collectivités ne se fasse pas départir de leur rôle dans l'Action logement de proximité. Madame la sénatrice, j'ai essayé de d'être vraiment totalement transparents, francs j'espère convaincante dans l'approche qui était la nôtre, vraiment je, je vous le dis avec la plus grande des sincérité, notre objectif n'est pas le casser les bailleurs sociaux, je, je le dis, je le répète et que tout ce qu'on propose tout ce qu'on propose, avec cette réforme, avec les 4 axes de la réforme que que j'ai indiqué tout ce qu'on propose aux bailleurs sociaux c'est discuter avec les bailleurs sociaux alors après l'effort qu'on leur demande si c'est c'est important parce que c'est ce cette modification à la fois du cadre financier à la fois du regroupement à la fois de plus d'accession sociale à la fois de participer à l'effort de diminution du modèle appel pour en assurer leur pérennité, oui, c'est un véritable effort, ça nécessite de choses que vous avez très justement rappelé, c'est prendre en compte les spécificités et prendre en compte la proximité, la politique de proximité, conseil, bailleurs sociaux, encore une fois, aujourd'hui un dans un débat avec les bailleurs sociaux, qui est que on part sur cet article 52 du projet de loi de finances, qui aujourd'hui sur la table, qui est la base de discussion, la base de de négociation que nous avons avec le je prends vraiment mot votre proposition de travailler avec les sénateurs, dans le cas de l'arrivée de cet article 52 au Sénat parce que, effectivement, toutes les discussions que nous avons amèneront je l'espère, parce que ça voudrait dire qu'on aura trouvé un accord entre nous tout ça à des modifications de cet article, dont il faudra qu'on discute ensemble, donc effectivement il faudra qu'on qu'on si discussion sur l'ANRU, on en reparlera également dans dans les autres questions mais je voulais vraiment insister sur ce ce on, la, la, la discussion notre volonté et la discussion qui est nécessaire et dans ces discussions évidemment au 1er jour, on a pris en compte leur contribution à à l'ANRU qui est un élément important parce que l'ANRU, ça peut pas être financée que par l'État, on le sait lire. Michel, ministre, la parole est à madame Annie Guillemot pour 2 minutes. 4,2 millions de logements HLM occupés par plus de 10 millions de personnes, 15 pourcent des des ménages qui relève du logement social, dont la moitié de ces ménages sont en dessous du seuil de pauvreté, avec un loyer moyen de 390 euros compte 570 dans le parc privé, les organismes HLM répondent à une demande sociale forte, d'autre part, comme nous le savons tous en cette assemblée, il gère au quotidien des grands ensembles qui souvent cumulé handicaps : chômage, dégradation de l'habitat, échec scolaire, délinquance sans l'implication de ces organismes HLM, quelles seraient les perspectives pour ces quartiers pour nos villes, compris dans les copropriétés privées dégradé où justement on va les chercher, non le logement n'est ni un luxe ni une marchandise comme une autre, le projet de loi de finances, prétend que les organismes HLM, dispose de 11 milliards de trésorerie dans les feuilles, dispose de 8 milliards en moyenne 10 et 2 mois d'activité, soit un ratio normal pour une entreprise saine, dont un 1000000000 de dépôt des garanties de locataires des provisions pour travaux planifiés, enfin, le résultat d'exploitation de 2 2 milliards est intégralement réinvestis dans la production et la rénovation du parc avec les effets du multiplicateur en termes d'activité d'emplois Directs et indirects des TVA à 800 millions dès leur parler, ne matelas ou de rentes relève de contresens l'examen attentif de l'article 52 s'avère mortifère pour le logement social, la baisse des APL revient à prélever aux organismes 1,7 milliards en 2018, 1,5 1000000000 en 2019 amputera leur capacité d'investissement de 75 pourcent une une ponction qui va diviser par 4 les opérations de rénovation et de construction neuve au détriment de Love, c'est pourquoi on peut pas vous suivant votre raisonnement en guise de contrepartie, le gouvernement propose un gel du taux du Livret A sur 2 ans, alors les organismes s'endettent sur 40 ans voire plus parler de contrepartie opérante et de leur hein leur plus d'une centaine d'organismes HLM vont être ainsi mis en péril, quand plus d'une centaine d'autres connaîtront les plus grandes difficultés présidés par des élus locaux, monsieur le ministre, des maires, vous semblez l'oublier je vais y venir vous ce sont généralement les villes qui garantisse la dette des organismes enfin, quel sera l'impact sur le financement de la rénovation urbaine, comme l'a dit ma collègue alors que les acteurs s'accordent pour estimer la note à 10 milliards d'euros, monsieur le ministre, alors que le logement est d'une cruelle activité, il serait plus raisonnable n'est-ce pas de surseoir à à l'application de l'article 2 du projet de finances. Pour 2018. on voit certainement les mêmes, mais je suis pas sûr que je vous dise exactement, tout est ce que ce que vous avez vu, mais je vais vous donner 3 exemples précisément est-ce que ce que vous, vous avez vu, vous disent : l'article 52 il s'appliquer en s'appliquant, ils ont, il a toutes les conséquences que vous évoquez très certainement est-ce que l'un d'entre c'est dit avec l'ensemble ce qu'appelle le package financier que je rêve, je réitère et tout à l'heure à la tribune, quels seront les impacts pour moi bailleurs je vous donner 3 exemples, il s'avère que dans le département du Rhône, je ne les nommerai pas, parce que dans le département de Rhône, vous avez aujourd'hui 3 organismes qui ont à peu près des taux d'autofinancement à hauteur de 15 pourcent,, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont à investir par rapport à l'ensemble de leurs fonds propres, ils vous disent vous disent : avec la réforme, moi je vais avoir aucune capacité d'autofinancement effectivement si vous prenez des 15, la réforme telle qu'elle est, elle, fait tomber ses 15 à 9 8 et 14 pourcent d'autofinancement en fonction des autres avec le package avec le package financier que nous proposons avec le paquet de avec le paquet financier que nous proposons, il s'avère qu'à chaque fois, vous revenez, revenez à hauteur de 12 et il y en a même un qui est à 15 qui passe à 17 pourcent de de capacité d'autofinancement la réforme avec le package lui-même bénéfique c'est ça, c'est ça la réalité, c'est-à-dire que on n'est pas encore une fois, on n'est pas dans cinq climat où on dit aux bailleurs sociaux, on va vous ponctionner de l'argent, on essaye, on essaye juste d'avoir une réflexion qui qui qui essaye d'être la plus intelligente possible certes, comme c'est l'État et la Caisse des dépôts, qui finance depuis 40 ans, sans jamais s'être posé la question mais comment on peut améliorer ce financement pourquoi depuis 40 ans fait que du taux variable et pas du tout fixe alors que ça fait un véritable gain pour en fait pas plus de près de haut de bilan, alors que c'est un véritable bien voyez pour l'un des officiers chez vous, le paquet de financer ça augmente même sa capacité d'autofinancement donc dans les critères comprend dans l'analyse comprend : il faut aller jusqu'au bout en prenant aussi les conséquences de l'amélioration du financement. Oui, Monsieur le Ministre, la parole est à monsieur Joël Guerriau pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors je voudrais saluer si l'initiative de mes collègues centristes qui ont mis au coeur de notre débat la question du logement social et on voit que dans la question finalement posée, se trouvent les des même de la diversité de nos territoires, un sujet qui mérite toute notre attention, nous manquons de logements sociaux pour des ménages qui peinent à se loger, c'est un constat : les derniers textes législatifs ont démontré que de louable dessein sur le papier pouvait aboutir sur le terrain à des objectifs inatteignables pour des territoires en capacité foncière et financière limitée ou conduisait à une offre inadaptée à la demande pour répondre aux objectifs de 25 pourcent de de logements sociaux, certaines intercommunalités ont intégré le principe de la mutualisation des objectifs trier nos de rattrapage des communes déficitaires dans leurs plans locaux de l'habitat pour atteinte de façon collégiale cet objectif à l'horizon 2025, quoi de plus naturel au sein des intercommunalités finalement une démarche incitative et vertueuse que la loi égalité et citoyenneté a failli supprimer un comble à l'heure où l'échelle de l'EPCI est désormais l'échelle privilégié des politiques d'habitat, d'urbanisme et surtout de déplacements urbains les les uns et les autres étant parfaitement liée avec la question du logement, alors que la charge du logement est aujourd'hui confiée au ministère de la cohésion des territoires et non plus à l'égalité des territoires, et ça c'est heureux : la mutualisation intercommunal permet la gestion des contradictions entre un objectif national uniforme et la prise en compte de la diversité des territoires et de leur histoire, ma question : pourquoi donc ne pas encourager la généralisation de la mutualisation des objectifs de logements sociaux au niveau des intercommunalités pour celles bien sûr qui le souhaitent et ainsi enclenché dynamique autrement plus positive que des amendes pénalisantes aux communes pour répondre au mieux, donc un enjeu Christiane, merci Monsieur miss. Merci, merci, merci pour le respect des 2 minutes d'ailleurs, monsieur le ministre, pour 2 minutes. Merci beaucoup monsieur le sénateur pour la question, donc, la question que vous posez renvoie plus généralement également à la question de l'application article 55 de la loi SRU

Aujourd'hui, au moment où on se parle, mais il faudra que on en discute avec vous dans le cas du projet de loi de logement que nous nous portons, c'est un débat que nous avons eue avec Jacques Mézard avec beaucoup d'autres, de savoir est-ce que oui ou non, il fallait qu'on touche à l'article 55 de la loi SRU, alors le sujet est très compliquée, parce que d'une part vous avez énormément de cas où quand on discute du cas c'est très justifié, c'est même ça relève souvent du bon sens, vous avez des communes, on sait très bien que si vous passez aussi vous laisser la loi telle qu'elle est, c'est mathématique, elles arriveront pas atteindre l'objectif de la loi, donc il y a même un effet démoralisant, c'est-à-dire qu'on nous dit ben on vous met un objectif mais on sait très bien, on sait tous ici que on n'arrivera pas à la fin, inversement, si vous indiquer que oui, on est prêt à ouvrir la loi SRU, en fait vous savez pas très bien comment la globalité va réagir quand j'ai la globalité, c'est l'ensemble, c'est-à-dire est-ce que si vous faites ça en si vous envoyez un signal en disant : la loi SRU, on en rediscute est-ce que à la fin. Vous ne craignez pas un manque de motivations de beaucoup, beaucoup sont très motivés, d'autres le sont un peu moins c'est c'est un euphémisme, et vous le savez bien, et est-ce que dans ce cas-là, vous créez pas en fait une reculade, dans la mesure où les gens se font sentir de moins en moins obligé par rapport à la loi SRU, c'est un vrai débat, il n'est pas du tout facile à trancher, à ce stade, on s'est dit que on ne mettait pas la loi SRU, dans le projet de loi logement mais le débat il est totalement légitime, moi, je rejoins votre question et il faudra que on en discute en préparation du du Merci monsieur le ministre, la parole est à monsieur Stéphane Ravier pour 2 minutes. Merci monsieur le président Monsieur minutes, permettez-moi de vous rapporter une tranche de vie, la scène se déroule au printemps 2014 dans le village de Saint-Marc, située dans le 7ème secteur de Marseille, qui compte 150000 habitants, dont 50 pourcent de de logements sociaux, le préfet de région, fait un point sur l'avancée des travaux de rénovation d'une cité sociale implanté dans le 14ème arrondissement, il a réuni, pour cela, le préfet délégué à l'égalité des chances, l'adjointe au maire de Marseille, en charge de la politique de la ville, appelons-là Arlette, un représentant de la police nationale et les bailleurs et le maire de secteur, récemment élu, en l'occurrence, votre serviteur seul pouvoir est absent, la presse, ce qui permet au préfet de nous annoncer directement et sans tabou, mais c'était sans compter sur le fait que je ne sais pas garder un secret, mesdames et messieurs, je suis très inquiet, l'objectif du programme est de recréer la mixité sociale, or nous allons droit à l'échec, c'est d'autant plus regrettable que ce programme est le plus coûteux : 180000 euros par logement, nous avons découvert dans cette cité et n'organisation clanique, les gitans ont chassé les Maghrébins, nous avons rencontré le chef des gitans, il est d'accord pour accueillir des familles qui viennent de l'extérieur, à la condition qu'elle soit gitane, nous nous sommes rendus ensuite sur les lieux et Arlette, l'adjoint de l'ONU, Jean-Claude Gaudin, de s'émouvoir et demain interrogé Stéphane, on ne va quand même pas laisser ces gens dans cette situation et de lui répondre humainement non et abandonnant un instant les versets de la religion laïque et obligatoire du vivre ensemble, Arlette, de constater et de nos confiés mais cela ne servira à rien, ou quand le mur de l'idéologie s'effondre

concentration des programmes sur les mêmes territoires communautarisme incivilités et insécurité qui interdisent à des familles d'accéder à des logements qu'elles ont financé et auxquelles elles ont droit et dont elles ont besoin d'émission et aveuglement idéologique des pouvoirs publics et se contente de les verser des sommes considérables sans aucun contrôle, sans aucune volonté d'y faire respecter, sinon le vivre-ensemble au moins le savoir vivre.

comptez-vous enfin tourner le dos à toute idéologie pour enfin prendre en compte la réalité des difficultés rencontrées par nos concitoyens dans les cités HLM. Merci, monsieur le sénateur, je je crois pouvoir dire avec fermeté que je ne partage absolument pas la vision, les propos que vous avez tenu tenu la conclusion de 2 de vos propos aujourd'hui c'est pas parce que on se dirait qu'il y en a qui sont plus prioritaires à d'autres dans les logements sociaux que vous allez régler quoi que ce soit de la situation que vous avez évoqué. La situation de la politique de la ville, on la connaît, ça fait 40 ans qu'on est dessus, ça fait 40 ans que les fractures, elle ne cesse de s'accroître, elle ne cesse de s'accroître, je suis pour ma part, absolument persuadé que c'est pas par le discours que vous venez de tenir qu'on va réussir à franchir ses frontières qui nous sépare des quartiers de la politique de la ville, en aucun cas, comment on fait pour avoir plus de mixité sociale parce que la vraie réalité, c'est que cette mixité sociale lutter contre ses frontières territoriales ses frontières de société, ça passe par des opérations de terrain très concrète, la, la, la plus forte qui qui était prise depuis des années, c'est très, c'est très certainement ce que nous venons de faire avec le doublement des classes dans les zones Red Très sincèrement, c'est une mesure qui aurait dû être fait depuis très longtemps qui était compliqué à faire, mais qui permet de donner un accès plus facile à l'éducation à à certaines personnes qui qui en ont besoin excusez-moi de pas répondre sur des critères d'attribution des logements sociaux, je pense très sincèrement que c'est un vecteur d'accroissement de ces fractures territoriales de divergences entre les sociétés plus qu'autre chose. chose. Ministre je rappelle aux collègues qu'ils ont 2 minutes maximum, donc il y en a qui ont très bien respecté ces 2 minutes. D'autres un peu moins, donc ce serait bien de pouvoir les respecter scrupuleusement donc je donne la parole à Madame Maryse Carrère voilà pour 2 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je risque d'être malheureusement redondante mais le département d'Hautes-Pyrénées n'échappe pas aux inquiétudes ressenties sur le territoire national sur ce thème, alors en matière de logement social article 52 a suscité de vives réactions de la part des bailleurs sociaux du département, et relève à mon avis d'une d'une vraie fausse bonne nouvelle pour les locataires, si l'État réalise par ce biais une économie substantielle au travers de la diminution du montant des APL, il n'en fait pas moins porter le poids sur les bureaux du budget des organismes HLM, mettant en péril leur équilibre financier et menaçant alors la qualité même des logements, certaines d'entre eux ont dores et déjà annoncé geler leur production de logements jusqu'à nouvel ordre, en effet, permettez-moi de vous donner l'exemple de l'impact que la baisse des loyers va aucun occasionné pour 2 organismes dans Les Hautes-Pyrénées tout d'abord, la société d'économie mixte de construction de la ville de Tarbes qui estime sa perte financière entre 500 et 600 1000 euros, se retrouvant avec un autofinancement négatif de 300000 euros l'OPH 65 évalue quant à lui cette perte à 4 millions d'euros, subissant une diminution de plus de 90 pourcent de de son auto financement des 2 organismes devraient alors faire appel pour leur encours alors garant qui ne sont autres que les communes et le conseil départemental dans la marge de manoeuvre budgétaire a été extrêmement mise à mal depuis plusieurs années, conséquemment à ses pertes budgétaires c'est d'habitat lui-même qui se verra amputé des programmes de rénovation et en particulier de la rénovation thermique ainsi lorsqu'à moyenne Tervel eut été envisageable de concevoir des économies liées à la performance énergétique du parc immobilier, l'absence d'investissement dans la matière, un gendre aura inévitablement des dépenses supplémentaires pour les locataires en fait cet article pourrait tout bonnement s'avérer aussi contre-productif pour atteindre l'objectif d'amélioration de l'accès au logement des personnes les plus modestes car en zone tendue particulièrement peut-on raisonnablement penser qu'au vu du danger financier que représentera pour un organisme HLM, le fait d'avoir une majorité de locataires pour lesquels il serait contraint d'abaisser les loyers, sa commission d'attribution continuera-t-elle à attribuer des logements aux plus modestes, cette démarche impliquant une diminution de ces retouches source monsieur le ministre. C'est beaucoup, madame la sénatrice tout à l'heure j'évoquais un office, une société qui pouvaient avoir jusqu'à même des impacts positifs avec les nouveaux modèles de financement, on l'art propose il y a un versement des offices ou des sociétés qui ont des impacts négatifs, vous avez raison, il y a là diverses. Et il y a 750 offices ou sociétés si on prend également les 5 ça monte à 800 le nombre d'entités aujourd'hui qui finance du logement social, vous le connaissez très bien, vous en avez tous et toutes sur votre territoire la difficulté effectivement, c'est un de réussir rapportés cette réforme du financement cette réforme de la vente, cette réforme du regroupement et, en même temps de réussir à faire en sorte que cette réforme que nous portons, elle n'impacte pas l'un qui est faible et et l'autre qui en serait ressorti encore plus fort, c'est une vraie, une vraie difficulté, alors dans l'article 52 il y a ce qu'on appelle une mutualisation une péréquation, chose que vous connaissez par coeur le travail que nous devons avoir dans la finalisation, c'est de s'assurer que cette mutualisation cette péréquation, elle est particulièrement pertinente : pourquoi tout à l'heure j'évoquais la TVA par exemple qui est une piste de travail que nous proposent les bailleurs sociaux, pourquoi c'est intéressant, enfin plutôt pourquoi ils préféreraient faire ces réformes avec un taux de TVA, tout simplement parce que le la TVA, ça c'est fonctions directement de votre activité, plus vous avez d'activité plus, vous pouvez bénéficier des financements nouveaux qu'on propose et plus en fait, vous utilisez ces financements nouveaux très attractif pour financer à moindre coût, votre nouvelle activité, vous voyez ce que je veux dire, et donc en fait, ça permet de faire une corrélation, indépendamment de l'impact et des structures financières des offices ou des sociétés aujourd'hui et donc ça, c'est un moyen d'avancer dans le bon sens, mais encore une fois, j'insiste, le ça n'est pas une décision budgétaire lampe le l'intérêt de diminuer les APL il est réel, il faut le il faut le faire parce que c'est la pérennité du système, mais c'est la réforme globale du système d'HLM qu'on essaie de porter aujourd'hui. Merci monsieur le ministre, la parole est à Madame, Dominique est trop si ça sonne pour 2 minutes. Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur la baisse des APL, puisque je vous ai posé la question dans les questions d'actualité, je parlerais plutôt de la politique du logement adapté à nos territoires et je regrette que la politique du logement du gouvernement s'inscrit dans une démarche interventionniste et centralisatrice, bousculant quelque peu les élus locaux et Racer resserrant l'étau autour des collectivités locales, le logement tout court, et plus particulièrement le logement social doivent répondre à une demande en fonction des territoires qu'ils soient tendu ou non dans les Alpes-Maritimes, par exemple en Île-de-France nos collectivités au nom des 25 pourcent de de logements sociaux d'ici 2025 se voit assigner des objectifs de production qui sont surréalistes et inatteignable en tout cas dans le délai imparti 2025 c'est demain ses obligations finissent par décourager les élus, même les plus volontaires dans la brochure de présentation de la stratégie logement du gouvernement, les collectivités sont loin d'être au coeur des dispositifs proposés alors que leur rôle central et d'initier localement une politique de l'habitat, au nom de l'intérêt général du principe de solidarité et surtout des spécificités des territoires, le maire, le maire de mer bien le 1er sollicité lorsque l'un de nos concitoyens, procède à une demande de logement social, il faut donner plus de souplesse à l'application de la loi SRU, non pas, comme je l'entends dire souvent pour exonérer les communes de leurs obligations de construction de logements, mais simplement pour permettre une meilleure adaptation des objectifs aux réalités des territoires, dans un souci de meilleure adéquation entre l'offre et la demande de logement, c'est la raison pour laquelle il serait plus pertinent peut-être de définir entre le préfet et les collectivités une contractualisation arrêtant les objectifs réellement réalisable au vu, par exemple, de l'état du foncier disponible des projets structurants définis et mise en oeuvre des sanctions s'appliqueraient à leur présence, la question cette contractualisation était pas respecté, alors Monsieur le Ministre, quel est votre avis sur cette adaptation aux réalités locales qui, je le pense sincèrement serait plus à même de créer un choc d'offre. plusieurs points le 1er point objectivement dans la politique du logement comporte avec Jacques Mézard, on a eu un souci des collectivités je vous donner quelques exemples, on a essayé

on va arrêter cette surenchère et on va passer sur des schémas de contractualisation avec les collectivités, c'est beaucoup plus efficace 2ème élément sur la loi SRU évoquais tout à l'heure, le débat, il est très compliqué parce que, objectivement, vous avez raison, il y a des approches territoriale l'exemple que vous avez donné c'est exactement celui que je prenais tout à l'heure, vous avez raison, vraiment la difficulté, c'est de se dire est-ce qu'on rouvre le débat plutôt si on rouvre le débat alors qu'il manque un 1000000 et demi de logements sociaux en France aujourd'hui est-ce que à la fin c'est contre-productif pour cette cause nationale qui doit être de faire plus de logement social, alors après il y a un 3ème point qui est la territorialisation de la politique de logement

c'est vachement bien pour territorialisée, une politique de logement, ça fait des années que ça dure, donc là on est en train de revoir cette territorialisation on va aménager les choses c'est de se dire comment cette fonction des différentes zones peut-être plus proche de la réalité, moi je pense qu'à terme, effectivement il faut territorialiser de plus en plus sa politique du logement, ça fait partie de ces politiques ou de faire la famille vient de l'Oise dans le petit village, vous avez pu de centre ville plus de centre bourg et en revanche énormément de pavillons autour, avec tous les problèmes que ça emporte chez les visiter un village analogue dans le Bas-Rhin, mais c'était l'inverse et pourtant les les 2 sont zone B2 et donc si on a les 2 dit on dit des financements des dispositifs qui ne permettent pas de faire la même politique, vous avez raison, et donc à terme il faut territorialiser ça prendra du temps en France. Michel, le ministre, la parole est à Monsieur André Gattolin pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mais question porte sur les entrées et les sorties dans le logement social ces dernières années, beaucoup a été fait pour favoriser la construction de logement social 9

notamment citer la TVA à taux réduit l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les avantages liés à l'accès à l'épargne réglementée et auprès locatif, si les objectifs initiaux du précédent gouvernement, ne sont pas remplies, la hausse du rythme de la construction, au cours de ces dernières années, doit nous réjouir néanmoins monsieur je veux porter bottes, attention, ce qui me paraît peut-être 2 écueils liés à cette politique du logement social centré sur la construction, il apparaît, d'une part que les constructions ne sont pas suffisamment ciblée et ne tiennent pas compte, par exemple, des zones de tension ou encore de la taille des foyers avec notamment l'accroissement des familles monoparentales, alors qu'on a des logements sociaux qui sont prévus pour un plus grand nombre de personnes, d'autre part, parmi l'ensemble des entrées dans le logement social, seule une sur 6 s'effectue dans du logement 9 dans une construction 9 alors comme la Cour des comptes, l'relevé la rotation au sein du parc social de morts aujourd'hui encore trop faible et il conviendrait, à mon avis utilement de favoriser celle-ci afin d'accroître le nombre global de logements proposés à la location sont tous focalisés sur la construction de logements nouveaux aussi Monsieur le Ministre, quels sont les instruments que vous comptez utiliser pour fluidifier les entrées et les sorties dans le parc social et au final est-ce qu'une plus grande fluidité ne permettrait pas à coût constant, une meilleure redistribution de la part des organismes de logement social vers les foyers aux revenus les plus modestes.

la question pour introduire plus de mobilité, elle est compliquée parce que et ça et ça rien d'ailleurs un peu la question de tout à l'heure, c'est c'est pas quelque chose qu'on peut décréter par une loi, c'est quelque chose qui soit au plus près du terrain et vous en êtes les premiers garants, tout simplement parce que. Les ménages qui constituent les logements sociaux, ils sont connus sur le terrain, on a fait comme je crois nous de porter un aménagement au niveau des commissions d'attribution des logements parce que ces commissions d'attribution des logements : elles sont composées de celles et ceux qui connaissent véritablement ce qui habitent dans les logements sociaux, notre objectif, c'est de pouvoir le faire sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on propose à celles et ceux qui habitent un autre logement tous les 6 ans si tant est que la situation familiale de ces derniers, que ce soit des enfants qui sont partis faire des études, que ce soit, inversement, un héritage qui leur a permis d'acquérir un appartement dans la rue voisine etc etc, de leur dire : on vous propose d'autres solutions et et si ces personnes à ont le droit au parc social, on leur propose d'autres solutions dans le parc social, et de toute manière, in fine, et on ne fait que leur proposer mais pourquoi il faut le faire rapidement, parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, aussi, quand vous avez, vous rentrez dans un logement social, faut qu'au bout de 25 ans, vos enfants partent de ce logement social ou plutôt que dans 25 ans votre bailleur social vous propose un nouvel appartement en fait l'évolution des prix est telle que votée 5, il a un loyer qui est inférieur à un T3 vous faites même pas de gains de pouvoir d'achat, donc vous avez juste aucun intérêt et donc vous arrive vous rester dans votre appartement, parce que ça ne vous intéresse pas, et vous avez bien raison de le faire et donc la question c'est de pouvoir le proposer suffisamment rapidement tous les 6 ans pour que soit un véritable gain de pouvoir d'achat pour vous. vous. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Fabien Guez pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'annonce était du coup de rabot sur l'APL a sonné comme un coup de tonnerre pour 6 millions et demi de foyers 5 auront à moins : c'est à moi de goûter pour les enfants ou encore les repas d'une journée comme en témoignait ce matin 2 bénéficiaires de l'APL dans le journal L'Humanité. Cette mesure injuste rapportera 390 millions d'euros au budget de l'État dans le même temps, Bruno Le Maire annoncé, nous allons rendre 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs à l'ISF en bref vous pénaliser les 20 pourcent des des ménages français qui ont le plus besoin d'aide pour se loger au profit des 1000 plus riches qui ont sans doute n'en ont pas besoin, il serait d'ailleurs intéressant de savoir s'ils appartiennent au 3250 familles qui dit selon Le Figaro du train de septembre dernier, 150 milliards d'euros dans les paradis fiscaux et vous allez encore plus loin en annonçant une baisse d'APL pour les locataires de logements sociaux, compensée par une baisse des loyers équivalentes, c'est donc aux bailleurs sociaux de compenser, encore une fois, le désengagement de l'État à hauteur de milliards 5 d'euros autant d'argent, moins pourrait les réhabilitations les constructions et le bien être des habitants, en fait, cette mesure crée une inégalité insupportable entre les locataires car demain les bailleurs ont plus de scrupules à loger des bénéficiaires d'APL dont les loyers seront plus faibles que ceux qui ne sont pas bénéficiaires de ces aides, d'autres personnes se verront barrer la route du logement social, car leurs revenus par seront en dessous du minimum requis par les commissions d'attribution, saisi par le collectif Vive l'APL, le Conseil d'État a promis qu'il rendrait sa décision avant vendredi, mais vous pouvez agir avant,

il y a plusieurs sujets le le décret dont vous parlez, c'est un décret d'exécution budgétaire sur l'année 2017 est-ce que c'était une bonne idée de raboter de 5 euros et ce que les politiques de rabot sont des bonnes idées, je pense que tout le monde sait suffisamment exprimé pour dire que c'est pas ça la solution,

défini et que cette diminution des APL, la presse, la mienne, la même montré, elle était déjà prévue maintenant c'est quoi la réforme si, si, mais si madame, je suis désolé mais enfin bon, on pourra y revenir, mais je suis désolé, c'est quoi, en revanche, les réformes que nous proposons, c'est la réforme actuelle, avec tous les débats qu'on a sur 2018 et ces mécanismes que nous essayons de mettre en 9 c'est-à-dire apporter des financements aux bailleurs sociaux permettez regroupement permette l'accession et en faire bénéficier le système notamment des appels pour en assurer leur pérennité et deuxièmement, c'est une autre réforme dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais il faudrait donc raconte dont on peut discuter si vous savez le l'établissement du revenu de vos appels sur quelle base aujourd'hui vous établissez vos APL, c'est sur la base des revenus est de. C'est pas vos revenus réels, c'est pas vos revenus actuels, donc quelqu'un qui travaille et il y a 2 ans et qui aujourd'hui est au chômage touche des appels au regard de son revenu il y a 2 ans, quand il était au travail avec un abattement forfaitaire qui fait mais qui ne correspond pas réellement à ses revenus du chômage actuel et ça typiquement, voyez, ça c'est une réforme qui est vraiment intelligente également dont personne ne parle, une réforme qui est beaucoup plus juste pour cette personne qui travaille, il y a 2 ans et qui, aujourd'hui, aujourd'hui, est au chômage et qui est aussi une mesure d'équité pour quelqu'un qui est au chômage, a 2 ans, qui est aujourd'hui au travail. J'le ministre, la parole est à monsieur Claude Kern pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, en propos liminaires j'insisterai sur le fait que la démarche, l'élaboration d'un projet de territoire en matière de logement qui soit social ou non, doit se faire en partenariat avec les collectivités locales, elle oblige à articuler la réflexion sur le logement au sein de son contexte territorial et de cette dynamique de développement et permet ainsi d'avancer de manière opérationnelle dans les territoires nous dispense disposant d'éléments pour prospectif Scott PLH Fradette entre autres, à ce titre, la montée en puissance des collectivités territoriales et de l'intercommunalité, ont eu un impact important sur les politiques du logement, or les contraintes sur les finances publiques devienne un des principaux sujets de préoccupation des acteurs dans ce contexte, il est primordial que les efforts soient maintenus, d'un point de vue fiscal en faveur des zones rurales pour soutenir les investissements immobiliers, en effet, le logement social ou plutôt aider un effet de levier particulièrement puissant, il constitue un investissement structurant pour les territoires alors opérer un réseau nage restrictif en matière de paix PTZ et de dispositif Pinel s'avère extrêmement contre-productif pour les territoires ruraux puisqu'on leur fait perdre en attractivité et on les fragilise encore davantage et ce ne sont pas les engagements du président de la République de prolonger de 2 ans, le PTZ neuf ou de 4 ans le PTZ ancien en zone B2, qui vont inverser la attente tendance durablement, et c'est la même chose en matière de taxation des plus values immobilières réalisées au moment de la vente de terrains, notamment le gouvernement propose comme le vous l'avez évoqué dans votre intervention préliminaire des dispositions dans les zones tendues tendue mais encore une fois, il ne faut pas oublier les territoires ruraux, pourquoi ne pas élargir ce type de mesure aux zones rurales et non tendues et jusqu'où êtes-vous prêt à aller le caser échéant par exemple exonération quand il s'agit de projets relatifs au logement aidé étant de réduction élevé pour les autres opérations je vous remercie pour les éléments que vous pourrez nous fournir à ce sujet, afin que nos territoires reste attractif en ce domaine et que les moyens développés puissent participer participer activement à la réduction de la fracture territoriale et sociale. Merci, monsieur le sénateur, plusieurs points 3 points très rapidement, l'importance des collectivités je répondais tout à l'heure à Madame national se hisse résister Hassan, un autre point que je n'ai pas évoqué, c'est pour ça par exemple, alors ça va mieux en le disant, puisqu'on ne le dit pas, nulle part dans notre stratégie indiqué, mais c'est pour ça qu'on a pris aussi un engagement très faire très ferme, pardon, de laisser, bien évidemment, le permis de construire dans la main des maires, sachant que beaucoup sont venus nous voir le 1er jour en nous disant : attendez la meilleure des solutions si on peut plus construire que soit du social, pas du social et autres, c'est surtout enlever le permis de construire dans la main des maires aujourd'hui vous construisez pas si l'élu local, il n'est pas d'accord, c'est pas vrai, donc on laisse bien évidemment le permis de construire dans la main des maires, ça va mieux en le disant, parce que souvent c'est quelque chose que qui est occulté sur les dispositif PTZ Epinal il faut aussi devoir voir de là on part en fait le projet de loi, les projets de loi de finances d'damant instaurer la fin de ce dispositif au 31 décembre 2017, tout s'arrêter partout, on a pris un engagement ferme de reconduire ce dispositif sur 4 ans dans la plupart des cas sur 2 ans, dans le 9 dans les zones B2 et C, je parle du PTZ 9 et de 4 ans dans ces mêmes zones sur l'ancien et pourquoi sur une aussi longue durée pour justement donner de la visibilité de la visibilité aux acteurs, mais aujourd'hui, objectivement, rares ont été les gouvernements qui ont pris un engagement d'or de rallonger sur une aussi longue durée ces instruments financiers, que ce soit en zone dense ou en zone détendue après la difficulté de détendu mais c'est tout l'enjeu de la territorialisation dès le début de la politique de logements aidés et des instruments, il y a des zones détendues, celle que j'évoquais tout à l'heure dans l'Oise où objectivement ce qui tue la âne du village, c'est d'avoir eu que des constructions aux alentours, par des dispositifs fiscaux et pas du tout de rénovation du centre ville, c'est pour ça qu'on va plus loin sur le PTZ ancien que le PTZ neuf dans certaines zones rurales, maintenant il y a des cas où l'exemple que je vous donne, il ne marche pas et donc aujourd'hui on fait comme ça, on fait au mieux, ça ça pose la question de la politique du logement à terme. La parole est à monsieur Joël Labbé pour 2 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Un aménagement équilibré des territoires en matière de logement social exige une répartition sur l'ensemble du territoire, de nouvelles constructions afin d'assurer à nos concitoyens de logement décent à des prix abordables, que ce soit en termes de location, mais aussi d'accession à la propriété dans la logique d'une stratégie contrainte par la diminution de la dépense publique, le gouvernement a fait le choix de recentrer le dispositif Pinel et prêt à taux 0 sur les zones tendues honni revient, cela va limiter forcément le développement des autres territoires en rajoutant des difficultés à monter des opérations mixtes logement social accession sociale accession libre en zone dite non tendues ainsi beaucoup d'intercommunalités vont se retrouver dans l'incapacité de mettre en oeuvre leur politique local sur l'habitat et notamment répondre à leurs obligations SRU ces mesures cumulées sont contraires aux attentes d'aménagement d'un aménagement équilibré du territoire, alors Monsieur le Ministre, une clé une question simple et très large, comment comptez-vous concilier ces 2 impératifs : faire face à la demande des zones tendues et accompagner les zones tendues dans le développement d'une attractivité attractivité renouvelé, je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, merci monsieur le sénateur, la, la, la question que vous posez, elle est au centre des débats que nous avions jusqu'à présent, c'est-à-dire la territoire territorialisation pardon à terme de toute la politique du logement, il y a certaines pistes, on sait que dans la zone, il faut construire plus, plus vite et moins cher, donc là c'est assez facile, vous faites le choc sur la fiscalité du foncier, vous faites un choc pour également dire aux entreprises chez tous les habitats que vous pouvez voir fait tous les locaux de commerciaux commerciaux, vous pouvez avoir pour construire des logements et et vous faites un choc également en reconduisant très fortement les dispositifs fiscaux permettant de construire sur ces zones-là avait quand même un souci, c'est de construire plus dense dans des zones pas très pas très dense pourtant tendu, on connaît trop ces ces exemples de bâti pas du tout dans son tour de gare en pleine métropole c'est un non-sens urbanistique et inversement, la question c'est que savoir comment on fait une politique d'aménagement du territoire, dans les zones détendues, l'exemple de dire sur le PTZ par exemple, on le croit conduit plus longuement sur l'ancien que sur le le 9 vise à répondre à cette problématique dire aujourd'hui globalement, globalement en zone détendue, il faut avoir un effort plus important sur la rénovation que sur la construction nouvelle, quand je dis ça je parle vraiment très globalement et j'aime pas vraiment de tels propos parce que, encore une fois et je pense que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, moi je suis convaincu que chaque territoire a sa spécificité et c'est très difficile de généraliser ces même le défi qui est le nôtre, voilà mais vous avez une question aujourd'hui des instruments qui existent, qui sont ce qu'ils sont et qui permettent que cette approche globale en revanche un dernier point que vous évoquiez, qui est l'attrait économique des territoires, moi j'ai passé des années à essayer de redresser des entreprises dans les territoires et je sais bien que l'attractivité d'un territoire, c'est pas que le logement c'est un triptyque : emploi, logement, transport, c'est pour ça qu'on essaye de pousser ses proies dans le même sens, mais ça renvoie aussi au plan de rénovation des villes moyennes que j'évoquais tout à l'heure où le volet économique très présent. Mon cher collègue, vous souhaitez impliqué, vous avez encore un peu de temps. Non, c'est bon, la parole est à Madame Viviane Artigalas je m'excuse parce que j'ai pas respecté l'ordre donc voilà, mais là quand même que 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ma question Monsieur le ministre concerne la baisse des APL, cette décision est injuste car elle va frapper en 1er lieu plus de 6 millions de ménages parmi les plus modestes et les plus précaires qui perdront 60 euros de pouvoir d'achat, chaque année, elle est injuste car elle devrait être compensée par une baisse des loyers HLM sans aucun Avantage pour les locataires, Paris, percussions, elle coûtera aux organismes HLM près de 1,7 1000000000 d'euros par an et les obligera à augmenter les loyers des locataires ne disposant pas d'APL via les surloyers, cette décision est aussi contre-productive, d'abord pour les offices HLM qui verront leur capacité d'investissement gravement compromise, que ce soit pour entretenir les bâtiments les rénover et en proposer de nouveaux avec la même qualité, les manifestations négatives de cette décision se font d'ailleurs déjà sentir en Midi-Pyrénées par exemple, ou 19 organismes de logement social, ont décidé de suspendre provisoirement le lancement de nouveaux programmes et toutes les opérations en vente en l'état futur d'achèvement, ces organismes n'auront pas d'autre choix que de recourir à la mobilisation des garanties d'emprunts accordées par les collectivités locales, ce qui les placera dans une situation fragile, c'est une mesure contre-productive contre-productive également pour l'activité économique du secteur du bâtiment qui peine déjà à se relancer, qui pourra s'en trouver fortement réduite, fragilisant ainsi la l'emploi local enfin telle allait contre-productive lorsqu'il s'agit de mettre en place et la transition énergétique décidée par le précédent gouvernement, en finançant notamment la rénovation thermique des bâtiments, monsieur le ministre, la politique du logement social et certes, certes, une question économique mais c'est aussi une question culturelle, nous vous parlons là d'un modèle de société que nous voulons avoir et nous voulons une société solidaire, vous n'ignorez pas que la décision du gouvernement un à la baisse des aides à la Pierre va fortement compromettre les réinvestissements des bailleurs et la construction de nouveaux logements sociaux dans le besoin se fait quotidiennement sentir dans nos territoires, alors ma caution est simple, monsieur le ministre attend réellement mesurer l'impact que cette mesure allait avoir sur l'économie locale, particulièrement particulièrement dans le secteur du bâtiment, nous soutenons de plus en France, le droit à des logements sociaux de qualité, comment allez-vous répondre à cette exigence avec une telle mesure.

toute la réforme ambitieuse que nous essayons de porter, elle est compliquée, elle est difficile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça nécessite beaucoup d'discussion et ça nécessite de prendre en compte toutes les inquiétudes, encore une fois, il faut être en revanche très juste, donc qu'on ce qu'on dit ou ce qu'on laisse dire sur le sujet, il s'agit pas, encore une fois d'aller ponctionner les bailleurs sociaux hétéro bailleurs sociaux ah ben, super, on va vous prendre un 1000000000 7 et ce sera dans les caisses de l'État, c'est pas du tout ça, qu'on propose encore une fois et j'espère en tout cas vous avoir montré tout tout tout ce tout ce qu'on proposait aujourd'hui aux bailleurs sociaux, y compris les évolutions récentes que nous avons fait, y compris des évolutions que nous ferons et je rebondis sur ce que disait la sénatrice Létard tout à l'heure, encore une fois, ces discussions, elles se poursuivront avec vous au Sénat dans le cas du PLF, je vous donne un exemple très concret qui englobe plusieurs points de votre question, on propose par exemple 3 milliards d'euros de prêt pour faire de la rénovation énergétique des prêts très avantageux, on propose en plus 600 millions d'euros d'un autre type de près encore plus avantageux, mais qui permet aussi de faire de la rénovation énergétique ces prêts sont faits par l'État, le coup le bénéfice de ses c'est-à-dire le l'Avantage la bonification comme on dit dans le secteur, c'est l'État qu'il prend à sa charge, à la fin ça permet quoi, ça permet de rénover, ça permet de faire une fini une diminution de coût des charges, on est bien d'accord, vous avez rénover énergétiquement donc vous diminuer les charges, ce qu'on dit nous simplement dans la réforme, c'est que l'objet social, la meilleure source d'un bailleur social c'est pas gagner d'argent, c'est pas de de garder l'argent c'est de plus construire et c'est de faire en sorte que cet argent qui l'argent des locataires soit investi la meilleure des façons hé ben si demain vous avez moins de charges à payer, quand vous êtes un office parce que c'est l'Office qui payent des charges, il en rétrocède une partie aux locataires, et si vous avez moins de charges à payer, de charges à payer, il est assez juste, que vous puissiez contribuer à améliorer un système, y compris dans son volet APL, voilà, c'est ça le raisonnement avec cet exemple très précis de énergétique avec les charges. Oui, monsieur le président, Monsieur le ministre, cette réforme du logement social et de l'APL préoccupe les bailleurs sociaux et les élus, et moi je suis assez surpris cet après-midi de la quasi-unanimité des propos, quels que soient les bancs dans cet hémicycle contre cette réforme, monsieur le ministre, ça a été dit, répété mais j'enfonce le clou : vous le savez bien moins d'investissement, c'est moins d'emplois pour nos entreprises locales.

c'est encore un risque supplémentaire que vous leur mettez sur le dos, et ça c'est une vraie inquiétude je voulais aussi vous vous dire ce sont des sommes considérables qui sont en jeu et des pertes financières énormes, où, à mon avis et je crois que c'est l'avis général, vos compensations promises ne seront certainement pas à la hauteur, vous ne voulez pas vous dites ruiné les bailleurs sociaux, alors merci de modifier votre votre ma 2ème question sera second point que je souhaite aborder sur les les difficultés d'application de la loi SRU, notamment dans les zones littorales, je suis en Charente-Maritime, où la politique foncière urbaine est strictement cadré. Chez moi une, une commune du littoral vient d'apprendre, par exemple la déprogrammation de 15 logements alors qu'elle doit rattraper un retard de construction, d'autres communes ont perdu leur droit de préemption au profit d'établissement public foncier qui peinent également réaliser des projets en raison du coût du foncier et du nombre d'agréments régionaux insuffisant, je pense également à la situation des communes nouvellement soumises aux obligations de construction de logements sociaux en dehors du zonage, il faut donc leur insertion des dispositifs d'aide, monsieur le Ministre envisagez-vous d'adapter les objectifs de construction territoire et quelle réponse : pouvez-vous apporter pour garantir une politique de l'habitat efficace. sur votre 1er point sur l'impact de l'article 52 je ne savais que redire avec insistance que ces impacts, il faut les entendre évidemment. Il faut les juger à l'aune de ce qui de ce qui est véritablement la réforme que nous proposons, et pas uniquement l'article 52 c'est l'ensemble des financements que je j'ai indiqué, c'est l'ensemble de la réforme sur le regroupement qui est porté par les offices et les sociétés elles-mêmes, c'est l'ensemble de ce que nous faisons sur l'accession sociale en discussion, hein, avec les offices et les sociétés, permettez-moi, par exemple, d'insister sur ce sur ce plan-là, je prenais tout à tout à l'heure, l'exemple des charges sur l'efficacité énergétique, ah c'est assez juste l'État finance l'efficacité énergétique et que les bailleurs sociaux peuvent le faire à moindre coût et qu'à la fin il et moins de charges à payer, qui puissent redistribuer ces charges c'est Seguin pardon et ne pas le garder que pour eux, mais de faire en en sorte que ce soit les béni des locataires qui en bénéficient tout à l'heure j'ai évoqué la vente accession sociale, j'ai indiqué que si on on ne vendait, ne serait-ce que 20000 logements à 100000 euros en prenant ce chiffre complètement par hasard, mais sur un parc de 4 1000005 ces 2 milliards de 2 milliards d'euros de recettes, soit à peu près 10 de l'ensemble des loyers versés chaque année, donc vous imaginez quel impact vous pouvez faire en diminuant le les loyers pour l'ensemble des locataires, j'ai même plus loin dans le département de Charente-Maritime, aujourd'hui vous avez 25000 logements sociaux. Vous avez 10000 demandeurs en attente 10000 et vous avez 2500 attribution chaque année simplement d'quand vous vendez par exemple en accession sociale un logement en moyenne faisant construisez 2 ou 3. donc la question fondamentale, c'est comment vous portez cette réforme d'ensemble, encore une fois, là elle est compliqué à faire parce que ça fait des années que le système fonctionne comme elle est compliqué à faire, mais il faut la portée in fine et. La parole est à monsieur Jacques Le Nay pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, samedi dernier, j'ai présidé l'assemblée générale de l'Association des maires et présidents de PC de mon département, les maires des communes périurbaines et rurales, mais également des communes insulaires ont rappelé avec insistance et difficultés rencontrées pour réponde besoin de logements en raison des règles d'urbanisme, c'est pourquoi, Monsieur le Ministre, me permettra d'appeler aujourd'hui votre attention sur les difficultés engendrées par la loi, allure l'impossibilité de construire dans Les Amours entraîne une situation catastrophique, tant pour les propriétaires que pour les personnes désirant accéder à un droit à construire, souvent des jeunes ménages dans l'espoir de bénéficier d'un prêt à taux 0 et bien entendu pour le tissu économique local, il ne faut pas se cacher derrière la protection des Terres agricoles pour justifier cette position dans la quasi-totalité des cas les donc re sont des bouts de jardin ou parcelles, la terre de terre à l'abandon au milieu des villages et hameaux totalement inadapté à l'agriculture, ces espaces représente à l'évidence à fort potentiel de foncier constructible disposant d'équipements et réseaux déjà financées par les communes, autre constat : dans le cas de la loi SRU, le mode de calcul pour le nombre de logements sociaux, Franck, on ne l'ensemble des résidences principales de la commune, au lieu de considérer le seul périmètre aggloméré ce principe de calcul communes étendue qui possède de nombreux écarts par corollaire 20 pourcent de de logements sociaux devient très difficile à atteindre, d'autant plus que ces communes se trouvent souvent éloignées du coeur de leur bassin de vie, compte tenu des difficultés qui s'annoncent pour les bailleurs sociaux, ces collectivités territoriales vont se retrouver doublement pénalisés, après 3 ans d'application de la loi, allure, le constat est sans appel : la grande majorité des maires souhaitent une évolution en urgence de certaines dispositions de cette loi pour honorer les objectifs fixés dans les PLH, alors Monsieur Mini-je voudrais savoir si vous pouvez envisager d'assouplir les dispositions de la loi allure rendant constructibles et donc creusant nos villages et hameaux, ce qui aurait pour effet d'éviter les nombreux contentieux dont font l'objet les maires de France, je vous remercie de votre attention. Merci, merci, cher collègue, rapporte monsieur le ministre, pour 2 minutes. Merci beaucoup monsieur le sénateur, vous avez raison il faut pas se toujours se cacher derrière des arguments, je suis ingénieur agronome, je sais bien ce que c'est que l'artificialisation des Terres agricoles mais premières amours et beaucoup de conviction, n'empêche que cette artificialisation des zones agricoles, vous l'avez pas au centre du hameau, comme vous l'avez évoqué les donc rose aujourd'hui, je parle sous votre contrôle la loi allure les permis déjà dès lors que, en fait, c'est déjà un bâti c'est pas que du foncier, c'est déjà un bâti donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez d'élargir sur du foncier, et pas uniquement sur du bâti. Aujourd'hui dans le projet de loi de logement qui est en cours de profs on n'avait pas identifié sujet donc on l'a, on l'avait pas évoquer maintenant avec grand plaisir d'en discuter avec vous, en en amont pour voir si on peut aller dans ce sens et et et en discuter le projet de loi de logement, on présentera en conseil des ministres mi-décembre et on le présentera au Parlement à partir du 1er trimestre 2018, donc on a encore un peu de temps devant nous pour pouvoir voir si il faut avancer dans dans ce sens. Merci monsieur le ministre, la parole est à monsieur Frank monte G pour 2 minutes. Chez le président, monsieur le ministre, chers collègues, le modèle économique du logement social France qui s'articule autour de 5 spécificité un équilibre financier à long terme, l'absence de bénéfices distribués loyer liée aux coûts de production, la transformation des dépôts sur livrets A un prêt à long terme, via la Caisse des dépôts et consignations et le recours à des subventions publiques, ce modèle est un fait tout d'une extrême cohérence il est technique et financier, il intègre la production et la gestion locative, il est basé sur les articulations du dispositif et ça, c'est le même public, aide à la personne et dans la Pierre et des prêts politique nationale et politique local et il repose sur la sécurisation systémique de tous les acteurs, y compris les locataires, compte tenu des décisions prises par le gouvernement sur la baisse des APL et l'obligation de baisse des loyers, la diminution des aides à la Pierre des conséquences des nouvelles règles du jeu de la fiscalité de l'épargne affectant déjà les dépôts des livrets A de l'augmentation des coûts de production, de logement et de l'affaiblissement des capacités d'intervention des collectivités, ce modèle et de fait remis en question, quel nouveau modèle parce que c'est de ça qu'il s'agit le gouvernement Hampton qu'il mettra 9 et sur la base de quel principe vous parlez vous-même de réforme, personnellement, je ne souhaite pas le changement de ce modèle, je pense au contraire qu'il faut le renforcer en donnant à tous les organismes HLM, le pouvoir effectif de répondre aux objectifs d'intérêt général fixé dans cette optique de justice sociale et d'égalité des territoires, et au regard de la diversité des situations financières constatées ne pensez-vous pas indispensable et urgent de mettre en oeuvre une péréquation nationale au bénéfice et des organismes les plus en difficulté souvent situés en zone rurale, mais pas seulement et se sentent dégradé la situation de ceux qui se portent bien, ou mieux.

je déteste les équilibres instables et autrement, c'est-à-dire que je pense que on avance plus vite on réforme plus vite en gardant un équilibre mais en voyant comment on peut améliorer cet équilibre, je vous donne un exemple très concret dans votre question, vous dites par exemple le taux du Livret A, c'est un bon élément pour le financement du du logement social, mais quand les taux sont très très bas, comme aujourd'hui, le Livret A coûte énormément d'argent aux bailleurs sociaux énormément, qui plus est, le taux du Livret A, il varie chaque année, ce qui, il faut pas le bailleur social et s'endette pas au taux du Livret A, ils s'endettent au taux du Livret A plus une marge la marche ça dépend quel est le type de logement mais cette marche, ça peut être jusqu'à ce en gros 1,1 ou 1,2 pourcent en en plus du taux du Livret A et donc dans un modèle comme aujourd'hui, vous avez des taux qui sont très très bas, pourquoi ce qu'on propose de faire des taux fixes avec un remboursement in fine, il est très intéressant par les bailleurs sociaux, parce que le taux du Livret A, avec cette marche très élevé pour les bailleurs sociaux aujourd'hui, donc moi ce que je dis, c'est qu'il faut garder les équilibres, mais en revanche comment vous améliorer ses ses équilibres avec par exemple cette fixation du Livret A pour donner de la visibilité de la visibilité avec, par exemple, c'est près de de long terme avec un taux fixé un remboursement est fini et puis 2ème point sur l'aide à la Pierre, moi, ma conviction, ça prendra du temps, on continuera à alimenter le FNAP mais le FNAP, on le sait bien, chaque année, vous avez le débat de savoir est ce qu'il faut mettre plus ou moins et on parle de 5 qui sont au final assez faible, la vraie discussion qu'on a avec les bailleurs sociaux aujourd'hui, c'est de se dire : si demain, si demain vous avez 8000 ventes aujourd'hui si demain vous passez à 20000 ou 30000 ventes passées vente en fait c'est des logements qui eux-mêmes avaient disposé d'une subvention de l'État qui avait disposé d'ailleurs de l'aide du FNAP hé ben, vous pourriez très bien dire que cette vente nouvelles à chaque fois il y a une partie qui va directement alimenter le Fnac et là pour recréer un système où, en fait, la vente finance elle-même la nouvelle construction si on arrive à faire un système vous pérenniser totalement le volet dans un équilibre au stade. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, comme d'autres collègues, je souhaite vous alerter sur le danger qui guette nos bailleurs sociaux qui n'auront plus la même capacité pour investir dans les territoires ruraux et notamment, dans mon département de la Mayenne, faute d'autofinancement en effet nos bailleurs sociaux Oruro ruraux vont être mis en grande difficulté par la contrainte des baisses de loyers qui va leur être appliquée, pourquoi, parce que nous avons un taux de d'appel Lisa Sion élevé avec de nombreux locataires à revenus très modestes et des loyers globalement à 15 pourcent en-dessous en-dessous des maxi autorisée et des loyers, qui sont aussi plus élevés ainsi avec le PLF 2018, nous aurons une baisse du loyer de moins 50 à moins 130 euros pour les locataires cette baisse imposée représente donc une perte de presque 7 millions d'euros pour les bailleurs sociaux de de mon département, ce qui est considérable, cela aura également un impact sur l'entretien du Patrimoine et les capacités d'accompagnement, un impact sur les entreprises du bâtiment et des travaux publics, dans mon département et bien sûr sur sur l'emploi local, l'impact également sur l'état, au travers de la TVA, mais les les grands perdants de ces mesures seront aussi les ménages eux- mêmes et en particulier les plus fragiles, les locataires du parc social, en particulier l'air un impact sur leur la modernisation de leur logement et c'est leur cadre de vie qu'il sera. Affecté alors Monsieur ministe, pourriez-vous nous préciser les contreparties à cette baisse de loyer, afin de permettre à nos bailleurs de continuer à investir, et je voudrais ajouter un mis ce qu'il faut bien tenir compte que les bailleurs sociaux dans les territoires ruraux sont souvent ceux qui permettent le lancement d'opérations privées Thierry toi et vous en avez évoqué notamment dans les centres bourgs, donc si vous voulez fragiliser vous obérer les possibilités d'opérations nouvelle donc dans ce domaine comme dans d'autres fait bien le discernement entre des territoires urbains et les territoires ruraux, je vous remercie. Merci monsieur le ministre. 3 milliards d'euros sur des prêts pour l'efficacité énergétique, la stabilisation du taux du Livret A à 2 milliards de reprennent de votre bilan 4 milliards d'euros de prêts à taux fixe, in fine, et 30 milliards d'euros de rallongement d'être 600 millions d'euros de prêt éco-PTZ voilà. tout ça c'est quand même une énorme manne financière maintenant la difficulté et le département que vous connaissez très bien en est un bon exemple, la difficulté c'est qu'effectivement le cas des offices sont très très différents et on sait je j'ai en tête un office sur votre territoire pour qui, effectivement, la situation est déjà complexe et des outils de financement qu'on propose ne lui sont pas forcément adaptées. On l'a en tête, on le connaît bien, et donc la question c'est : comment vous faites vis-à-vis d'Intel bailleurs de faire en sorte que ce c'est-à-dire j'évoquais un un office qui est une société qui elle aurait même un gain positif, comment vous faites pour vous assurer qu'à la fin il y a une mutualisation une péréquation et que vous ne retrouviez pas dans un cas où un office. Pourrait être significativement impacter alors que d'autres en tirer uniquement profit donc ça, on a bien en tête, ça serait par de la mutualisation ma péréquation et par une organisation entre les acteurs, donc ça se discute en ce moment avec le mais lequel vous l'âge auquel on a déjà en tête. monsieur le ministre, la parole est à Jean Claude Tissot. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2018 le prêt à taux 0 pour la construction de logements neufs et supprimé dans les zones dites non tendues sur les zones B2 et C,

le montant maximal du prêt à taux 0 accordée aux ruraux ne pourra pas dépasser 20 pourcent de de l'emprunt total compte 40 pourcent aujourd'hui aujourd'hui renchérir ainsi le coût de l'accession à la propriété pour les ménages modestes dans les zones rurales aura des effets non souhaitables, les familles les plus modestes, de l'acquisition d'une construction neuve ramener ces familles qui souhaitent investir dans le 9, dans les villes qui souffrent déjà d'une concentration de personnes à faibles ressources à contrario des efforts de mixité sociale. Et enfin mettre en difficulté l'artisanat et l'économie locale hors des grands centres urbains et d'ailleurs vous n'avez pas répondu à la question de ma collègue à ce sujet-là, sur ce point précis, bien Artigalas tout à l'heure, j'espère que j'aurai une réponse claire sur ce point là, d'autre part, nous constatons dans nos communes que les bailleurs sociaux ne veulent plus investir dans les territoires ruraux, de fait, le manque d'investissement dans le parc HLM des zones rurales, commence à se faire sentir durement, il devient ainsi indispensable de rénover les bâtiments construits dans les années 90 Nombre de ces logements sont de véritables passoires énergétiques engendrant des chars, engendrant des charges parfois supérieurs aux loyers l'APL, même diminué perd ainsi beaucoup de son sens qu'elle n'a pas, ils ne portent que sur le loyer, les bailleurs sociaux ne peuvent ni effectuer les investissements nécessaires ni s'en séparer pour des raisons comptables aussi je souhaite proposer des pistes à explorer pour leur permettre de transmettre leur Patrimoine en zone rurale sans aggraver leurs difficultés actuelles pourrait-on par exemple envisager un dispositif par lequel serait faciliter l'acquisition de ces bâtiments par les communes souhaitant revitaliser leur et mener des programmes sociaux, dans le cadre de la stratégie de logement du gouvernement, il est prévu de faciliter l'accession de locataires à la propriété en sécurisant l'achat-vente grâce à une structure dédiée, c'est cette structure viseraient à simplifier et multiplier le nombre de ventes à l'occupant à moyen terme, portant le nombre de ventes à 40000 logements par an, nous exprimons nous préciser ce dispositif, je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le sénateur, alors il y a beaucoup beaucoup de questions dans votre question, j'ai commencé par la dernière sur le le dispositif en question aujourd'hui, vous avez. Pour faciliter l'accession sociale et je parle vraiment d'accession sociale hein, pas du tout de la vente à des institutionnels et qui plus est privée, vous avez plusieurs sujets : vous avez un certain nombre de mécanismes qu'on peut simplifier parce que c'est vrai que ça relève aujourd'hui un peu du parcours du combattant, quand vous êtes un office et que vous voulez faire de l'accession sociale, donc dans le projet de loi logement et il faut qu'on ne y travaille tous ensemble, toutes les idées sont sont bonnes à prendre pour faciliter et puis après vous avez un 2ème sujet qui le sujet de la copropriété, les bailleurs sociaux aujourd'hui, c'est un euphémisme, et vous le connaissez par coeur, si je dis qu'ils ne sont pas totalement fan de la copropriété et on peut le comprendre, c'est pas leur métier d'être copropriétaire, c'est pas leur métier et donc comment on fait pour, mais comment on fait pour améliorer cette copropriété, donc là aussi dans le projet de loi logement on essaiera d'améliorer ce dispositif mais la structure dont on parle, c'est une structure qu'on a discuté avec Action logement avec l'USH sociale de l'habitat, de savoir est-ce qu'on pourrait pas imaginer une structure qui rachèterait schématiquement des immeubles directement et cette structure, elle, elle, elle se elle sort gérer la copropriété parce que ce serait sa finalité que de gérer de la copropriété et donc c'est ça l'idée, c'est d'une structure qui pourrait, en mais pour les bailleurs qui le souhaiteraient bien entendu racheter directement le bloc, si je puis dire pourri gérer directement la copropriété puisque certains ne sont pas fans sur le 2ème sur le 2ème volet sur les prêts à taux 0 dans le 9 en zone rurale, effectivement, diminue cette quantité alors cette quotité on a diminué après beaucoup de discussions avec les parties prenantes, c'est pas une quantité qu'on a inventé en sortant de de notre chapeau et vous les aurait remarqué qu'on ne la diminue pas dans l'ancien, c'est toute la problématique qui répond une partie de votre question, de savoir comment pour revitaliser plutôt que vous reconstruisait en 9, c'est un vrai sujet et donc l'outil PTZ ancien versus PTZ 9 en zone B2 et C, est un outil aussi d'aménagement du territoire compliqués avec des effets collatéraux mais on a essayé de bien calibrée. Le ministre, la parole est à monsieur Antoine Lefèvre. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le rôle des bailleurs sociaux sur nos villes moyennes et sur nos centres bourgs est déterminant et vous le savez, Monsieur le Ministre, avec une production annuelle de 230 logements 90 logements démolis et 50 vendues aux locataires l'office HLM de l'année, de langues que je préside encore il y a quelques jours, est un acteur local indispensable surmonter victoire 200 logements réhabilités thermiquement par an, 50 millions d'investissement annuel, plus de 500 emplois non délocalisables notre bailleur local revitalise nos centres bourg en transformant les anciens bâtiments publics en reconverti sont friches en construisant des logements adaptés aux seniors près des commerces et des équipements, la promotion privée n'est pas là pour le faire, car le marché n'est pas sur notre territoire les très gros bailleurs HLM ne s'intéresse qu'on métropole régionale, seuls les bailleurs locaux permettent de moderniser l'habitat de laine de façon visible ne doivent pas devenir des agences locales de gros bailleurs HLM lointain mais tout à l'heure dans votre réponse, vous nous avez dit que l'objectif était bien de favoriser les grosses office pourtant, la France doit enrayer une dynamique de fracture, fracture territoriale très engagée sur un territoire comme seuls les bailleurs locaux répondent à cet appel : comment, Monsieur le Ministre, avait voulu proposer une loi qui peut réduire à néant la capacité d'investir de HLM comment Monsieur, le ministre avait voulu proposer une loi sans mesurer ni simuler les conséquences sur notre territoire, la réduction de loyer de solidarité que vous souhaitez imposée aux bailleurs sociaux pour compenser la baisse des APL va transformer un office HLM, ça en a l'office HLM déficitaire sur nos nos fils, ce sont plus de 6 millions d'euros par an, le voilà déficitaire rendu par vos mesures incapable d'investir, monsieur le ministre vous proposer des compensations très flou à ce jour, elles sont pour la plupart inadapté pour nos territoires fragiles et prioritaire de fait vous nous demandez de voter un projet de loi de finances pour l'article 52 relatifs au logement social n'ait pas abouti dans son analyse des risques vous exposer ainsi les collectivités qui ont garanti les emprunts des bailleurs que votre projet de loi rend déficitaire et donc concrètement en situation de mettre en jeu, c'est garanti, je vous invite, comme l'a d'ailleurs très bien fait, Daniel Dubois dans son introduction à repousser cette mesure et je vous invite également à prendre le temps, le temps de prendre des tops testez vos mesures sur notre fils afin d'entériner une loi nuisible dans sa formule actuelle pour la cohésion de nos territoires cohésion à laquelle pourtant, nous savons par ailleurs attaché, je vous remercie. Dans votre département dans le sur le département de que vous représentez, il s'avère que, il y a une activité qui est peut-être beaucoup plus performante que dans beaucoup d'autres territoires, je vous donne un exemple concret : vous avez un nombre de logements sociaux, qui a 40000 aujourd'hui, il y a à peu près 5000 demandes et il y a chaque année 3000 attributions, ceux qui sont des ratios qui sont vraiment dans la fourchette la plus haute de ce qu'on peut connaître sur tout le territoire et donc tout ce que vous venez de dire : vous avez tout à fait raison, il ne faut surtout pas casser une dynamique, surtout sur des territoires comme le vôtre où ça marche, ça pourrait marcher mieux ça marche pas toujours marche mieux, et encore une fois, il y a quand même 2000 personnes qui chaque année n'ont pas accès au logement social, mais il n'empêche que ça marche quand même déjà bien en tout cas beaucoup mieux que sur d'autres territoires je vous donner l'un exemple très concret, en fait, vous avez un office, une société qui est en perpétuelle activité vous l'avez bien redit dans votre question, c'est pour ça tout à l'heure là puisqu'on évoqué et que monsieur sénateur du mois également dans son propos introductif de la TVA piste qui est une piste intéressante, notamment pour des offices ou des sociétés d'HLM comme celle de votre territoire parce que objectivement tous les financements que j'ai, vous avez dit qu'ils sont un peu flous, je n'en suis pas sûr qu'il soit flou, ils peuvent être difficiles à appréhender, mais ils sont pas du tout flou et en plus ils ont fait l'objet de communication très précis avec l'ensemble des bailleurs sociaux, mais c'est vrai que, ils sont d'autant plus favorable aux offices, qui sont dans l'activité, or la TVA était aussi un vecteur d'activité, c'est pour ça que les offices et les sociétés non voici travailler avec dans ce moment sur la TVA parce que l'un est très compatible avec l'autre, donc vous voyez cette situation que vous décrivez, on l'a vraiment on en discute et on aura l'occasion d'en discuter au Sénat avec. Merci monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jean-Raymond Hugonet. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, mes chers collègues, la loi SRU est un texte complexe qui a modifié en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement en France son article le plus notoire L article 55 qui impose aux communes de plus de 3500 habitants 1500 en Île-de-France, de disposer de 25 ou 20 pourcent dans dans certains cas, de logements sociaux à l'horizon 2025, cette loi appliquée de manière comptable et dogmatique, soulève des difficultés aussi ainsi certaines communes ayant fait le choix de l'intercommunalité ou se trouvant dans l'obligation de le faire, à la suite de la réforme territoriale se retrouvent contraints d'appliquer les taux de logements sociaux obligatoires, alors que ces derniers sont manifestement inadaptée à la réalité du territoire essentiellement composé de Bourg d'un habitat majoritairement pavillonnaire et encore éloigné de bassins d'emploi. La question du logement social doit s'apprécier sur un territoire donné de manière globale, certaines communes possèdent peu de terrains constructibles, elles peuvent à l'inverse, avoir sur leur territoire des espaces naturels protégés ou des zones d'intérêt patrimonial remarquables. Il semblerait donc logique que les injonctions faite aux communes et communautés d'agglomération pour réaliser des logements sociaux prennent en compte ces espaces spécifiques en minorant d'autant le taux obligatoire de logements sociaux aussi, je souhaiterais savoir quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour établir une analyse objective des besoins et capacités réelles des communes afin d'éviter des coupures d'urbanisation sur des zones présentant un intérêt sur le plan environnemental et paysager, on ne peut à la fois vouloir préserver un territoire de l'urbanisation dans un texte, et prétendre imposer une urbanisation dans un autre les 2 s'appliquant en même temps à un même territoire, ne pourrait-on pas plutôt apprécié les efforts réalisés par les communes, au regard des contraintes réelles et de ne pas se contenter d'un examen exclusivement comptable des logements construits, merci de votre attention. Merci beaucoup monsieur le sénateur, c'est un débat qu'on a évoqué à plusieurs reprises ici si vous prenez votre territoire il y a peu près 110000 logements aujourd'hui sociaux aujourd'hui, chaque année on en attribue 6000 le nombre de demandeurs 30 2000. Donc ça veut dire que, il y a un manque à peu près d'un quart, il faudrait avoir un quart de plus de logements sociaux dans dans sur notre territoire et donc la la difficulté, encore une fois, moi je l'entends, mais totalement hein et et en répondant tout à l'heure sur l'artificialisation des sols, j'ai fait toute ma formation et dedans je et dedans je général Gronholm je je je je connais par coeur ce sujet, la difficulté c'est que il y a des zones où il faut densifier, on sait qu'il faut densifier, construire une maison autour d'une gare en terme urbanistique, c'est aberrant, c'est d'ailleurs un des objets du Grand Paris, il faut pas construire des petits pavillons autour des gares du Grand Paris, il faut construire des vrais projets d'urbanisation forte, dense, parce que vous avez le tramway et le métro qui qui arrive et dans d'autres zones de se dire on relâche la pression, la difficulté c'est quand vous voyez que sur 110000 personnes, vous en avez 30 2000, qui sont en attente d'un logement, mais la difficulté c'est que si vous relâcher l'attention dessus vous mettez quand même beaucoup de personnes sur le bord de la touche alors qu'ils en ont besoin, donc encore une fois. Idéalement, vous avez raison il faudrait réussir à territorialiser au maximum, évidemment la question qui se pose à nous tous, et alors qu'on appelle déficit est-ce qu'on ouvre ce chantier avec un risque de dire à tout le monde en fait, on peut être cool sur l'atteinte de ces Jeux, objectif alors qu'au même moment, vous avez autant de personnes en attente, à ce stade, on a dit qu'on n'y touchez pas, le projet de loi n'a pas de composante SRU, on aura le débat dans les chambres, évidemment avec.

nous sommes pas de la même sensibilité, mais nous ne voulons pas pour autant votre échec je ne suis pas constructif mais je suis positif et j'ai surtout envie que notre pays réussissent alors j'ai entendu vos réponses aux nombreuses interrogations de mes collègues qui sont aussi, d'ailleurs les miennes mais alors que notre débat prend fin, je ne comprends toujours pas votre politique, vous voulez : d'un côté et construire des logements rénovés, le Patrimoine et en même temps vous baissez les moyens financiers des organismes sociaux, avec toutes les conséquences déjà longuement évoqué non seulement je trouve ça démagogique, mais c'est surtout une une catastrophe pour nos communes parce que votre politique va inévitablement, même si vous voulez vous forcer les bailleurs sociaux à faire jouer les garanties d'emprunt que les communes leur ont accordé en cascade, encore une nouvelle fois mettent les communes en difficulté et nos locataires, puisque c'est eux qui sont au au coeur de ce de ce sujet du logement, hé bien ils ne vont plus bénéficier des travaux d'entretien de réhabilitation de rénovation et ça, c'est une véritable catastrophe, alors oui la la cohérence dans tout ça, je je m'interrogeais un peu le sentiment quand même que vous êtes en train de vouloir assassiner des offices publics en pensant là qu'il y a comme une espèce de trésor caché, ce qui n'est absolument pas le cas, et puis surtout on évoquait tout à l'heure si vous voulez absolument que les Offices du logement social, vous savez qu'il faut dans le même temps, reconstitué, or les offices de pour reconstituer ce Patrimoine qui, s'ils en ont les moyens financiers et donc si on leur coupe leurs moyens financiers, mais ne pourront pas le faire et donc votre politique

Monsieur le Ministre, moi j'ai besoin que vous nous rassuriez de façon claire, pourquoi voulez-vous remettre en cause un système de de financement qui fonctionnait bien jusqu'à présent, et puis une 2ème petite question rapidement sur les attributions de logements, qui mieux que le maire, qui est mieux placé que le maire pour attribuer le logement or dans la loi précédente, on a fait en sorte que ce sommet dans le préfet qui rétribue sans connaissance des lieux sans connaissance de la cage d'escalier, les attributions de logements, il faut que vous fassiez confiance aux élus, je pense que vous l'air de de les estimer les porter dans votre coeur, même si vous n'avez peut-être pas été vous-même, il faut redonner aux élus locaux, cette possibilité, ce pouvoir d'attribuer les logements sociaux. Monsieur le ministre. Merci beaucoup et puis je profite de ma dernière prise de parole pour vous remercier toutes et tous ceux de de ce débat, oui, j'ai essayé d'être rassurant mais en parlant avec beaucoup de franchise beaucoup de conviction, j'ai essayé de vous expliquer de manière didactique, quel était le sens de la réforme que nous portons, quels étaient les éléments que nous proposions aux uns et aux autres et quel était notre boussole qui était de faire en sorte que aucun locataire allocataires ne puisse être pénalisé, bien au contraire, de répondre à une attente d'un 1000000 et demi de ménages qui aujourd'hui n'ont pas accès au au logement social, quelle est la politique si on devait la résumée en une phrase, uniquement une phrase sera forcément trop courte, concise mais trop courte, moi j'ai l'intime conviction que le système aujourd'hui qui ne repose que sur les APL, mais c'est un système qui est pas pérenne, donc on a le choix : l'évoquer dans mes propos introductif qui il a 40 ans, on a fait ce choix de la pub de l'aide personnelle au logement aujourd'hui, c'est une erreur 18 milliards d'euros chaque année c'était 14 il y a quelques années, ça en sera 24 prochainement mais c'est pas tenable, on peut dire ce qu'on veut quand les aides personnelles au logement alors qu'en même temps, représente la moitié du du budget de la défense nationale, alors qu'en même temps vous avez un Français sur 6 qui se considèrent en étant déficience de logement c'est pas tenable, donc il faut réformer le système en étant moins dépendant des APL et en trouvant des systèmes plus juste, plus innovant en améliorant les financements en favorisant l'accession qui permet de plus construire qui permet également d'alimenter l'aide à la construction, qui permet en plus de faire ce parcours résidentiel, c'est une telle approche en rénovant énergétiquement les bâtiments si une telle approche qui à la fin nous permet d'être moins dépendant d'un système qui continue inexorablement à à augmenter ce système des APL pour arriver à un système beaucoup plus pérenne et qui soit un système qui permette in fine et de construire plus au bénéfice du 1000000 et demi voilà, c'est ça la logique, c'est difficile, c'est difficile, ça était beaucoup plus sain de ne pas le faire, c'est difficile, ça n'est pas une logique purement budgétaire, certes il y a ce volet budgétaire puisque les appels dérive mais ça n'est pas ça, ce que nous essayons, ça n'est pas uniquement ça, loin de là et j'espère vous avoir convaincu, c'est de pouvoir changer, inverser la tendance est au promettre le système dans le bon sens en alignant les intérêts comme je n'tout à l'heure. Merci, mes chers collègues, le le débat sur le logement social est donc terminé, je remercie Monsieur le Ministre, de sa disponibilité et de ces réponses, nous allons passer donc lors du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d'eau potable Monsieur par messieurs Bernard Delcros et René Vandières, une banque et plusieurs de leurs collègues à la demande du groupe de l'Union centriste. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Bernard Delcros, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes.

Bien Madame la la ministre. Monsieur le président de la Commission, monsieur le président, monsieur le rapporteur de la commission, monsieur le président de séance, pardon mesdames, messieurs, mes chers collègues. Tout Hollande demande parcours d'élu local. Comme maire d'un tout petit village du Cantal et président d'une intercommunalité rurale, j'ai pu mesurer combien au fil des ans. L'accumulation d'obligation de démarches en tout genre de réglementation de procédure. à complexifier la tâche des élus locaux. Et parfois pénalise les territoires et tout particulièrement dans les petites collectivités qui ne disposent pas des équipes, des services techniques ou administratives pour faire face à ses obligations subit. Parmi l'ensemble de ses obligations. Certaines sont bien entendu nécessaires et c'est le rôle de Viel, des élus, de les mettre en oeuvre, mais pour d'autres leur empilement, les laissant parfois inopérante incompréhensible, voire contradictoires ou inefficaces. Je pense donc que, tout en veillant à accompagner les nécessaires mutations environnemental et sociétal, nous devons aussi avoir le souci permanent de simplifier. De clarifier d'alléger les procédures, c'est aussi je pense un gage d'efficacité. Je pense que c'est possible dans de nombreux domaines, sans faire de grandes révolutions mais par des mesures simples, pragmatiques, des mesures concrètes qui correspondent aux réalités du terrain. C'est précisément l'objet de la proposition de loi que je vous soumets aujourd'hui au nom de la délégation aux collectivités territoriales et la décentralisation que préside notre collègue Jean-Marie Bockel, j'y reviendrai tout à l'heure, de quoi s'agit-il. La simplification que je vous propose concerne le service public de distribution d'eau potable. Qu'ils soient gérées par la collectivité compétente en régie ou confier à un délégataire. Il s'agit de simplifier la procédure de déclaration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et d'éviter que les collectivités subissent à tort une pénalité financière. Pas une petite pénalité par le doublement de la redevance. Qu'en est-il aujourd'hui au cours d'une même année, les collectivités sont soumis à une double obligation. Une première avant le 1er avril, date à laquelle elles doivent transmettre à l'Agence de l'eau, la déclaration pour prélèvement sur la ressource en eau. Faisant apparaître les indicateurs de performance de l'année, un oiseau. Et c'est à partir de cette déclaration. Fondée sur des données non consolidées. Que les agences calcule le montant de la redevance et applique éventuellement le doublement de cette redevance et les indicateurs de performance ne répondent pas un certain nombre de critères fixés par l'agence poursuivant. Après cette première déclaration d'avril arrive la 2ème obligation, celle de 37 ans. Par laquelle les collectivités doivent publier le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, ce qu'on appelle le RP QS cette fois avec des données consolidées et tant pis pour les collectivités qui aura été pénalisé indument. Voilà donc une situation incompréhensible pour les collectivités qui sont contraints de communiquer les mêmes indicateurs performance 2 fois par an, à quelques mois d'intervalle en avril puis en septembre, il faut couronner le tout. Pour couronner le tout, à cette situation, s'ajoute une autre incohérence pour les collectivités qui ont délégué la gestion à un tiers le délégataire est tenu de fournir à la collectivité compétente les données consolidées nécessaire à la déclaration d'avril n'ont pas avant le 1er avril mais avant le 1er juin. Cette majoration n'est pas anecdotique. Le Conseil national d'évaluation des normes estime qu'elle représente environ 15 pourcent du du coût global des majorations. On voit bien que cette situation est aberrante et le dispositif inefficace. Le Conseil national d'évaluation des normes évalue le surcoût. Cette majoration abusive, si je peux dire à environ 520000 euros, Vise tout simplement à rectifier cette incohérence de date à simplifier la procédure déclaration et à protéger les collectivités d'un doublement de la redevance comment. L'article 1 il vise à empêcher le doublement à tort du taux de la redevance, du fait de donner non consolidé avant le 1er avril enfants dans la déclaration de la redevance sur les indicateurs de performance, non pas de l'année, de moins en mai de l'année N donc finalement. à partir des données consolidées, qui ont été publiées dans le rapport. De septembre précédent, donc de l'année moins ainsi le surcoût annuel de 528000 euros que j'évoquais tout à l'heure serait. L'article 2 attentats à rapprocher des obligations déclaratives existant en imposant aux agences de l'eau de près remplir la déclaration. De redevances d'avril puisque les agences disposeront des éléments pour le faire, à partir du rapport qui ont été présenté le 30 septembre de l'année précédente, ainsi les collectivités aurait à fournir leurs indicateurs performance une seule fois à l'occasion de la présentation du rapport en septembre. Enfin, l'article 3 propose la suspension pendant 2 ans du doublement du taux de la redevance, quelles que soient les indicateurs de performance constatée. Ainsi ce doublement ne serait pas appliquée en 2020 et en 2021. Pour les les manquements constatés en 2018 et en 2019, ce qui offrirait aux collectivités une période de transition sécurisé sans majoration de redevance et puis l'article IV propose l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2020, je sais que la commission ajuster un peu le texte pour permettre à l'Outre-mer, de bénéficier de ce que le dispositif qui suit évidemment extrêmement favorable pour terminer, je tiens quand même à rappeler l'origine de cette proposition de loi, elle s'inscrit dans le cadre de la mission de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, une mission qui a été confiée à la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, par un arrêté du bureau du Sénat de novembre 2014. Un sujet sur lequel notre ami et collègue Rémy-Cointreau en charge du dossier à la délégation est très investi essai inscrit aussi dans la charte de partenariat signé en avril 2016. Par le président Larché par Alain Lambert, le président du Conseil national d'évaluation des normes et Jean-Marie Bockel, le président de la délégation cette charte a pour objet de favoriser les synergies entre la délégation et le conseil et le conseil national d'évaluation des normes pour un plus efficace notre action en faveur de cette simplification des normes et c'est dans ce cadre que le Conseil national d'évaluation des normes a saisi le 1er février 2017 notre délégation qui a bien voulu me confier d'abord confiée à René Vandierendonck, que je salue au passage, qui a fait le choix de ne pas se représenter aux élections sénatoriales et à moi-même le soin d'élaborer cette proposition de loi et afin d'aboutir à une proposition partagée, nous avons souhaité établir un maximum de concertation avec l'ensemble des partenaires concernés et nous avons organisé le 20 juin dernier une table ronde, parmi lesquels, bien sûr, le Conseil national, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et le ministère de la transition écologique et solidaire je dois dire que, en fait un travail approfondi, nous avons eu de nombreux échanges au cours, c'est-à-dire, tables rondes et par la suite, ce qui a permis d'aboutir à une solution équilibrée qui est appuyée aujourd'hui, je pense par l'ensemble des acteurs de ce sujet, je veux remercier vraiment l'ensemble des participants et des partenaires pour à la fois leur engagement et leur esprit d'ouverture qui a permis de trouver une solution, celle que je propose, aujourd'hui, je vous invite donc, mais, chers collègues, à donner une suite opérationnel, c'est ça qui compte ou au final, c'est que ça puisse devenir opérationnel qu'on puisse appliquer cette mesure simplification à la province être position et je vous a remercie par avance. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pierre, le rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la ministre, cher collègue, sommes réunit aujourd'hui pour discuter de la proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d'eau potable. Cette proposition était déposée, vous l'avez entendu par nos collègues, Bernard Bernard Delcros, René Vandierendonck, le 1er août 2017 elle a été cosignée par plusieurs membres de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Il s'agit aussi d'une initiative transpartisane démarche que je salue cette proposition de loi permet de répondre à un problème bien identifié dans le domaine du service public d'eau potable qui a été soumis au sénat en application du partenariat conclu le 23 juin 2009 16 ans, pour le président du Sénat Gérard Larcher, le président de la délégation le président de la délégation aux collectivités territoriales, Jean-Marie Bockel, et le président du Conseil national d'évaluation des normes notre ancienne collègue Albert Lambert. Chargé de répondre à cette saisine, ne collègues : Bernard Delcros et René Vandierendonck ont mené une importante travail de concertation avec les différentes parties prenantes avant d'élaborer ce texte, je tiens à les saluer pour la justesse et le pragmatisme de leurs propositions. En effet, ce texte propose une solution concrète à des difficultés administratives réelles rencontrées par de nombreux élus locaux, il s'agit, en substance, donc problème de calendrier pour la transmission de certains indicateurs qui conduit parfois à une majoration indue de la redevance pour les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable. En décollant donnons la transmission de ces indicateurs, le texte permettra une application stable du mécanisme de majoration par ailleurs en prévoyant le pré-remplissage par l'Agence de l'eau de la déclaration effectuée avant le 1er avril à partir des éléments transmis au préalable dans le cadre du rapport sur le prix et la qualité de service, il réduira également la charge administrative imposée aux élus locaux. Cette initiative parlementaire illustre parfaitement le rôle constitutionnel du Sénat, de représentants des collectivités territoriales. Elle témoigne aussi de notre engagement en faveur de la simplification des normes qui s'appuient depuis plusieurs années sur une mission spécifique particulièrement active, dirigé par notre collègue Rémi pointeront au sein de la délégation aux collectivités territoriales. Enfin, ce texte concrétise le partenariat établi avec le Conseil national d'évaluation des normes en ce sens, il montre la voie à suivre pour, je l'espère, de nombreuses autres initiatives de simplification dans les prochaines années, nous en avons grand besoin. Tout commence au manteau commissions qui adopté cette proposition de loi à l'unanimité, il faut le souligner, je vous proposerai de la soutenir sans réserve. Nous ferons ainsi oeuvre utile en faveur des collectivités territoriales. Permettez-moi de conclure en évoquant de façon plus globale à la question de l'eau dans nos territoires, la qualité de l'eau nécessite une attention permanente, à la fois pour assurer l'alimentation en eau potable, mais également pour le lutter contre les pollutions et pour préserver les écosystèmes. La réduction des contaminations résultant de l'usage de pesticides ce sujet de d'actualité ou de certains Anglais doit être une priorité en identifiant dissolution du restitution pour nous agriculteurs. Par ailleurs, dans les prochaines années, la ressource va devenir de plus en plus rare et précieuse.

Il est indispensable de poursuivre nos actions pour réduire ses pertes à l'avenir, la gestion de l'eau devra permettre de mieux la préserver et de résoudre les conflits d'usages qui vont se multiplier, au-delà du présent texte nous devons donc être très vigilants et actifs sur ce sujet afin d'assurer une utilisation raisonnée équitable et durable de ces biens communs, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre, l'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, chère Claire mais deviennent mesdames et sénatrices, messieurs les sénateurs. C'est une proposition de loi innovante qui nous réunit aujourd'hui grâce à l'initiative de Bernard Delcros de l'ancien sénateur été vous avez salué René Vandierendonck et je tiens tout particulièrement à les remercier, proposition de loi qui est innovante dans sa genèse et que monsieur le rapporteur, vous avez présenté des collectivités ont alerté le Conseil national d'évaluation des normes de difficultés administratives, un diagnostic qui a été effectuée et il est apparu nécessaire de faire évoluer la loi grâce à un partenariat conclu entre ce conseil et le Sénat, les parlementaires ont pu trouver une solution en réunissant ensemble en réunissant l'ensemble des acteurs concernés, les collectivités et les représentants de l'État et tout ça dans un délai finalement assez bref parce que la saisine initiale du Conseil par les collectivités ne remonte qu'à quelques mois. Et ce processus ministre parfaitement la logique transpartisane qui doit nous guider, nous guider pour améliorer l'efficacité collective de nos institutions et nous guider aussi pour rechercher la simplification Guénot mécanismes administratifs et des mécanismes, il sera dit que le gouvernement met en oeuvre et l'empilement d'ailleurs que vous avez rappelé ici bien expliquer, du haut de votre expérience d'élu local, Monsieur le Président et monsieur le rapporteur, et donc en l'espèce, cette méthode à trouver à s'appliquer aux mécanismes de déclaration par les collectivités des informations nécessaires au calcul des redevances des agences de l'eau, en particulier pour la mise en oeuvre d'un dispositif de doublement de la relevant de la redevance pour prélèvement d'eau pour l'usage au potable lorsque certaines conditions de diagnostic ou de rendement des réseaux ne sont pas réunies. L'application de ce dispositif d'incitation fiscale des collectivités à faire des économies d'eau bien qu'essentielles à l'arrêt à la rénovation, nos réseaux distribution il s'est en effet avéré avéré administrativement complexe à l'usage, et cela pèse particulièrement comme vous l'avez bien souligné aussi et à plusieurs reprises, monsieur le rapporteur, ça pèse particulièrement sur les collectivités locales et donc la solution consiste à décaler d'un an, la majoration de la redevance pour donner le temps nécessaire aux collectivités pour transmettre aux agences de l'eau, les données techniques nécessaires au calcul ça permet d'éviter ainsi l'émission de titres de redevances majorées donnant lieu à des rectifications, ainsi que des surcharges administratives inutiles. Enfin, cette proposition de loi permet aussi une bonne application du principe, dites-le nous une fois en permettant aux agences de l'eau, d'utiliser des informations déjà transmises par les collectivités dans un autre cadre. Je tiens donc à remercier à nouveau les parlementaires qui ont su écouter les acteurs concernés et trouver une solution équilibrée qui, tout en préservant l'esprit des textes et en permettant la poursuite de la modernisation de nos réseaux. Simplifie le travail des collectivités sans aggraver la charge de travail pour nos agences de l'eau, celle-ci effectuant depuis plusieurs années un effort de maîtrise de leurs effectifs. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le gouvernement soutiendra cette proposition de loi, ensuite la proposition d'extension de la simplification aux offices de l'eau des départements d'outre-mer. Je défendrai simplement 3 amendements rédactionnels qui vise à améliorer encore sa lisibilité et donc à faciliter son application par les agences et fils de l'eau et leur redevables.

Monsieur le Président, Madame le secrétaire d'État, cette proposition de loi technique vise à répondre à un problème concret des collectivités en effet sont parfois amenés à subir indument une majoration des redevances sur l'eau, ce qui ne sont pas souhaitables dans le cas de la baisse continue des dotations fort que nous formulons cependant plusieurs réserves, premièrement si la simplification proposée constitue un progrès réel pour les collectivités qui n'auront plus qu'une seule déclaration à remplir, il s'agit cependant d'un transfert de chars lourds de de charges lourd pour les agences de l'eau. Celles-ci devront développer les techniques informatiques et former des personnels pour remplir leurs nouvelles missions. Or la situation des agences de l'eau étendu puisqu'elles verront leurs moyens financiers et humains réduire dans le cas de la loi de finances pour 2018. Une telle situation, aura des conséquences écologiques et économiques au détriment de la gestion patrimoniale des réseaux d'eau et d'assainissement. Deuxièmement, en gage de stabilité pour les collectivités, la majoration du taux de la redevance liée à un mauvais entretien ne serait pas appliquée ne serait si les collectivités ne vous vous ne doivent pas être inutilement pénalisés nous considérons nécessaire de prendre en compte l'état des réseaux dans la souci d'incitation à la Prévert, préservation de la ressource. Un mot plus particulier celles sur les territoires de montagne, le prélèvement sur la ressource est parfois plus important que ce qui serait nécessaire, cette situation héritée d'aménagement anciens a permis par le versement de trop plein d'eau, de créer une biodiversité particulière ces communes de montagne sont taxés inutilement alors qu'il n'est pas souhaitable de modifier ce fonctionnement cette situation mériterait aussi une réglementation adaptée. Pour finir, il convient de lier les difficultés des collectivités à fournir les éléments aux agences de l'eau à alors père globale de savoir-faire dans ce domaine, il ne convient donc pas d'agir uniquement sur l'allégement des normes, mais également de leur apporter un vrai accompagnement de leur mission de service public de l'eau, cet accompagnement doit se réaliser à travers une structure nationale dotée d'un corps de fonctionnaires formés, cela est indispensable pour remplir auprès des élus locaux, les missions de conseil mais également pour profiter promouvoir une utilisation économe de la ressource, il est inacceptable et dangereuse que l'expertise se situe quasiment exclusivement au sein des majors de l'eau de la même manière, à force de complexité de réglementation mal adapté, comme par exemple les transferts automatiques de compétence, de nombreuses collectivités vont être amenés à faire le choix de la délégation de service si nous sommes donc favorables à la simplification des normes Cécile ne doivent pas se faire au détriment d'un service public de qualité, la situation actuelle des agences de l'eau nous paraît beaucoup trop fragile pour la rajouter une nouvelle charge et donc pour ces raisons, nous observons nous abstiendrons sur ce texte. Merci, Merci, cher collègue, la parole est à Alain Madame, Nelly Tocqueville pour le groupe socialiste, vous disposez de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la Commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre assemblée donc examiné, aujourd'hui, cette proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d'eau potable, celle-ci a été déposé au Sénat le 1er rôle dernier par vous, Monsieur, velcro et notre ancien collègue René donc je salue ainsi que les membres auxquels je me suis associé de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, ce qui témoigne particulièrement du caractère transpartisan de celle-ci, cette PPL est l'aboutissement de travaux menés en amont au sein de cette délégation sur la simplification des normes, en effet, elle s'inscrit dans la continuité de la signature, le 23 juin 2016 d'une charte de partenariat entre le Sénat et le Conseil national d'évaluation des normes dont l'objectif principal consiste à mettre en avant une simplification des normes applicables aux collectivités territoriales et notamment donc aux dispositions législatives afférentes aux services publics d'eau potable, c'est la raison pour laquelle le CNN a saisi le 1er février 2017 la délégation collectivités territoriales sur ce point, afin d'examiner l'origine des difficultés rencontrées par l'ensemble des acteurs comme PCI mais aussi les agences de l'eau, cette proposition de loi, hé bien le fruit, nous pouvons le vérifier la riche travail de concertation avec ceci et le ministère de la transition écologique et solidaire, par ailleurs, une table ronde portant sur ce même objectif c'est tenu au Sénat le 20 juin dernier la difficulté majeure mise en avant par le CNN résulte de l'articulation de 2 obligations auxquelles sont assujetties les collectivités territoriales, à savoir d'une part, l'obligation pour celle-ci de devoir enseigner les indicateurs de performance tels que celui du rendement du réseau ou encore de la gestion du Patrimoine devant figurer dans la déclaration de la redevance pour l'usage d'alimentation en eau potable avant le premier avril de l'année suivant celle où le montant et du et, d'autre part, l'obligation pour le maire d'une commune où le président d'un EPCI de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, devant le conseil municipal où l'assemblée délibérante permettant de consolider ces mêmes indicateurs et ce avant le 37 ans, le caractère précoce de la date du 1er avril peut en effet amené des collectivités, a déclaré des données non consolidées, alors que le rapport rendu au 30 septembre permet quant à lui, de renseigner des indicateurs de façon plus, en outre, il est nécessaire de signaler que cette situation oblige les collectivités a effectué 2 opérations de relevés d'informations, ce qui engendre en conséquence des coûts supplémentaires, la proposition de loi sénatoriale que nous examinons, a pour objet de mettre en oeuvre, je cite, la solution de simplification équilibré et opérationnelle répondant aux difficultés des collectivités territoriales, sans désorganiser toutefois les agences de l'eau et en particulier en l'espèce, afin que les collectivités n'est plus à supporter de surcoût, elle permet par ailleurs que le mécanisme de doublement de taux de la redevance pour une année se base sur les indicateurs de performance de l'année, M. moins 2 et non pas de l'année, M. moins hein, ainsi on s'assure que ceux-ci sont bien consolidé, il faut également salué la mesure visant à suspendre temporairement de façon transitoire en attendant la mise en oeuvre effective des dispositions prévues aux articles 1 et 2 la majoration du taux de la redevance, alimentation en eau potable pour les prélèvements effectués en 2019 ainsi qu'en 2020, date à laquelle le présentoir entrera en vigueur, il est important de noter que cette proposition de loi a reçu un accord de tous les acteurs concernés, notamment les agences de l'eau, et cela même alors que celle-ci, il faut le souligner subiront une légère baisse de leurs recettes en conséquence notre groupe votera cette proposition de loi, je le rappelle, adopté à l'unanimité en commission au Sénat, car elle va dans le bon au sens et remplit pleinement l'objectif fixé, que nous nous sommes donnés de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Alain Fouché pour le groupe, les indépendants et pour 3 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, chats, collègues, vous le savez la loi notre entraîné une importante redistribution des compétences de nos collectivités territoriales, ces transferts de compétences ne se sont pas toujours fait sans douleur faute parfois un manque de concertation et à une baisse conséquente des dotations afférentes à ses compétences perdues aujourd'hui de nombreuses collectivités sont surchargés, du poids de nouvelles responsabilités sans pour autant être accompagné financièrement dans ses obligations, il s'agit de la question de la compétence au exercé jusqu'ici par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, le texte portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoyait son transfert obligatoire aux EPCI au plus tard le 1er janvier 2020, le Sénat, à la demande des maires l'avaient rejeté à l'unanimité en début d'année, toutefois, l'Assemblée nationale renouvelée à réintégrer cette obligation, il y a quelques jours, les territoires n'ont une nouvelle fois pas été écouté aujourd'hui la législation impose aux communes et EPCI le versement d'une redevance annuelle sur les prélèvements en eau de leur territoire, cette situation entraîne un calcul par anticipation de la consommation des collectivités territoriales, le caractère approximatif des estimations, c'est que les communes PC y sont régulièrement soumis, Madame la Ministre, à des opérations de régularisation, voire à des pénalités financières imprévisible et coûteuse pour leur budget, par ailleurs, le contexte financier des collectivités que chacun de nous connaît nous oblige plus que jamais à leur donner la visibilité nécessaire à la gestion des Budgets communaux soucieux d'accompagner nos communes et EPCI dans une simplification de leur démarche et obligations administratives, le groupe des indépendants ne peut que s'associer à cette démarche de simplification des normes et d'assouplissement de la législation mais, chers collègues, le territoire attendent des mesures fortes, écoutons-les, je rappelle que j'avais à ce propos, déposée il y a quelques mois, une proposition de loi précisant qu'une norme nouvelle adoptée devait en faire disparaître une existante, il perd, elle finira par venir un jour, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Olivier Léonard pour le groupe RDSE et vous disposez de 3 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la Commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est tout d'abord comme sénateurs nouvellement élu que je tenais à m'exprimer pour la première fois dans notre assemblée sur cette proposition de loi qui incarne parfaitement les actions de bon sens qui doivent, me semble-t-il, être porté par le Sénat, ce type d'initiative essentielle pour le quotidien de nos collectivités doit être multipliés pour renforcer l'efficacité et la crédibilité de notre action publique et donc la vitalité démocratique de notre pays n'ayant pas pu participer aux travaux préparatoires sur ce texte, je voudrais saluer la démarche partenariale le travail mené par les collègues qui ont suivi ce processus pragmatique et transpartisan jusqu'à aujourd'hui, on se focalise, bien souvent sur le trop de normes en matière de simplification, mais ce texte, c'est aussi l'occasion de rappeler l'enjeu de l'amélioration des normes existantes et il reste beaucoup à faire, je ne reviendrai pas en détail ici sur le bien-fondé de chacune des dispositions prévues mais je souhaite en revanche insister sur les conséquences indirectes de cette mesure qui pourrait apparaître au premier abord purement technique et sur ses bienfaits concrets dans la gestion du bien public, de l'eau, j'ai moi-même dans les précédentes fonctions comme maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, président de coeur des San agglomération territoire de 200000 habitants en région parisienne, conduit le passage, une délégation de service public, de 10 communes avec 10 contrats distincts vers une régie publique de distribution d'eau potable, ce n'était pas un choix idéologique mais une décision pragmatique transpartisane dans un territoire avec ses spécificités pour assurer un service public qui garantit aux usagers une eau de qualité optimale au juste coût, or si nous agissons aujourd'hui pour que les redevances et les majorations les majorations appliquée par l'Agence de l'eau soit fondée sur des données consolidées, il faut souligner que cette mesure participera indirectement à renforcer la connaissance des réseaux de distribution et donc de rationaliser les choix d'investissement pour éviter les pertes et les gâchis d'eau en simplifiant le fonctionnement du service public d'eau potable, nous encourageons notre collectivités à s'investir plus avant un sa gestion du quotidien nous Ankara encourageons donc des investisseurs manque plus pertinents par une meilleure connaissance des réseaux et nous participons donc à et diminuer les pertes d'eau car il faut être clair : les opérateurs qui vendent l'eau n'ont pas toujours eu intérêt à parfaire leur connaissance des réseaux de distribution, et il s'avère souvent difficile, voire impossible de connaître avec précision le rendement des réseaux de distribution à l'échelle de tout un territoire ou d'un secteur lorsque les bassins desservis par les producteurs d'eau s'étendent sur des surfaces bien plus vaste, c'est notamment le cas en région parisienne, il nous faut donc développer des outils de mesure précis du rendement des réseaux, la reprise de la distribution d'eau potable par les régies publiques doit s'accompagner de l'installation de compteurs sectoriel qui permettent des investissements optimisé avec un impact certes certain sur le coût de l'eau et donc sur leur pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, avec ce texte, au-delà même de notre volonté de simplifier basé les majorations de l'Agence de l'eau sur des indicateurs fille able, nous participons à réduire ces majorations en tant que telle, par une meilleure gestion du bien public, de l'autre,

Monsieur le Président, Madame la Ministre sur rapporte mais sa collègue, c'est devenu une habitude pour nous, nous avons une nouvelle fois, parler de la question de l'eau, transfert de compétences des limitations de celle-ci. Restauration des continuités écologiques, financement des agences de l'eau, composition des instances de Bassem, sans oublier les inévitables fuites d'eau sur le réseau d'eau potable ou même les contraintes d'autorisation de pompage, les occasions pour nous de se saisir des questions afférentes à l'eau ont été nombreuses malheureusement devant l'instabilité législative et financière devant les libertés d'interprétation COS autorise parfois, l'administration, les élus locaux se trouvent désemparés et c'est souvent sur le Sénat qu'ils concentrent leurs espoirs, cette proposition de loi et donc nouvelle lustration du rôle et du devoir de notre assemblée, celui de se porter au chevet des collectivités locales et des élus qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe en haut. Je voudrais d'abord saluer le travail patient de nos collègues : Bernard Delcros Piermay deviennent et Jean-Marie Bockel, certains considéreront sans doute que sa portée est assez modeste, mais je préfère un petit pas une idée générale qui produit une loi incolore et insipide. Dès lors, cette simplification constitue une réponse concrète apportée au syndicat des eaux aux collectivités locales qui prouvent, généralement les plus grandes difficultés à fournir des indicateurs de performance consolidée, il s'agit donc de permettre aux communes de déclarer les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource anneaux qui est assis sur le volume d'eau prélevés au cours d'une année si la transmission ni les éléments est au 1er, ravi de l'année suivante, alors même que la présentation du RP QS 37 tambour de cette même année, il n'y a rien d'étonnant à ce que les élus et des difficultés, a déclaré des données consolidées, le Conseil national des normes a même évalué l'économie à 500 même cumul Euro c'est peut-être modeste mais ça suffit, me semble-t-il, a justifié l'intervention du législateur, un mot sur le financement quand même des agences de l'eau car madame la ministre, vous le savez, l'État a pris la mauvaise habitude d'imputer chaque année, le fonds de roulement des agences de l'eau, ça 75 millions d'euros cette année. depuis 2013, c'est une habitude régulière autour de sa millions d'euros, tout cela pour financer son propre budget. Ce prélèvement plutôt cette captation, sans compter une diminution drastique et imposer des effectifs, de ce point de vue, le projet de loi de finances prochain prévoit une fois de plus, de piétiner le principe que je croyais sacro-sainte de l'eau paye l'eau, qui cherche à notre ami Rémy-Cointreau et ce qui inévitablement pénalisera, par contre, les Claude activités locales et syndicats qui les agences de l'eau travailler qui réduira par conséquent leur capacité d'intervention s'agissant d'incompétence, j'ai ma petite-fille de ses contours, il conviendrait que le gouvernement clarifie sa position sur le traitement des eaux pluviales, je rappelle que le Conseil d'État et ne ressentent circulaire nous indique que cette compétence relève du bloc j'aime, alors que le code des collectivités locales, nous indique le contraire malgré ces perspectives difficiles, je me réjouis que le Sénat prenne ses responsabilités, que nous puissions adopter cette proposition de loi, j'espère que le gouvernement assumera ses responsabilités et usera des outils que lui seul a à sa disposition, je vous remercie.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je suis ravi, moi aussi, jeune élu de prendre la parole aujourd'hui dans cet hémicycle pour défendre un texte qui réunit quasiment l'ensemble des formations politiques du Sénat, il s'agit, là, vous en conviendrez, d'une situation qu'il nous faut apprécier achat juste valeur ce texte empreint de pragmatisme de bon sens, formule une solution concrète à des difficultés administratives réels que connaissent nos communes, partout en France, en métropole, mais aussi chez nos amis ultramarins au nom du groupe La République en marche, je salue l'objectif de simplification portés par cette proposition de loi transpartisane l'intense travail d'évaluation et de concertation réalisé tout au long de ces derniers mois, ainsi que l'investissement des rédacteurs du texte et de notre rapporteur, la simplification, vous le savez, est un combat de tous les jours et ce sujet a d'ailleurs été évoqué lors du débat organisé ici même hier sur l'aménagement du territoire et je suis persuadé que nous aurons l'occasion d'y revenir encore et encore, cette simplification et s'inscrit pleinement dans le cap fixé par le président de la République lors de la conférence des territoires et le gouvernement ne doute d'ailleurs qu'elle sera parmi d'autres sujets au coeur du congrès de l'Association des maires de France de novembre prochain, avec cette proposition, mes chers collègues, nous nous engageons bien volontiers sur cette voie et faisant ainsi, avec cette proposition de loi que nous avons adopté ce soir figure de 1er de cordée, j'en profite, en ce sens pour également salué le partenariat signé entre le Sénat et le Conseil national d'évaluation des normes en 2016. Parti du réel de nos territoires et de nos communes, cette proposition de loi permet de lutter concrètement contre une insécurité financière vécue par un grand nombre d'élus locaux, ça a été rappelé, cette mesure de bon sens supprimera le risque de majorations indues à l'obligation de transmettre des informations à une échéance trop précoce et réduire à une charge administrative non négligeable qui pèse sur nos communes au plus proche des problématiques, des territoires, le Sénat est ici pleinement dans son rôle de représentant des collectivités territoriales et j'en suis heureux une fois adoptée en cette fin de journée, je formule dessous et le 1er que cette proposition de loi soit rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et le 2ème que ce texte transpartisan en faveur de la simplification pour nos territoires et nos entreprises, soit le 1er d'une longue liste qui nous permettra ainsi de partir du réel pour tendre vers un idéal, celui de l'efficacité au service des politiques publiques et de nos concitoyens pour toutes ces raisons, bien évidemment, le groupe la République en marche votera ce texte. Merci, Merci, cher collègue Monsieur Jean-François Longeau pour le groupe Union centriste dispose de 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la ministre mis chers collègues. La présente proposition de loi n'est pas seulement consensuel, elle est aussi technique et c'est un texte important, je ne dis pas cela uniquement parce qu'il est inscrit dans l'espace du groupe UC auquel j'appartiens. Ni parce que son auteur et notre collègue Bernard Bec velcro que je félicite au passage si ce texte est important, c'est parce que la méthode ayant présidé à sa génère devient devrait inspirer l'ensemble de nos travaux, une véritable concertation, une véritable démarche de simplification, et un résultat transpartisan, le tout sous la houlette de notre délégation aux collectivités territoriales c'est cela qui devrait être la marque de fabrique du Sénat. Je ne m'étendrai pas longuement sur le fond, l'objet du texte en effet déjà été très bien exposé par notre collègue permet de Viel, dont je salue au niveau au nom du groupe Union centriste l'excellence du travail surtout dans des délais aussi contre. Le texte simplifie les rapports entre les collectivités, les agences de l'eau dans le cas de la redevance sur les prélèvements en euros sur 2 points : d'une part aujourd'hui pour déterminer le montant de la redevance due au titre d'une année, chaque collectivité doit transmettre avant le 1er avril de l'année suivante, les volumes prélevés ainsi que plusieurs indicateurs de performance, ces déclarations avant le 1er avril pose des difficultés à bon nombres de collectivités qui ne disposent pas donné pas donné aussi tôt dans l'année pour remédier la proposition de loi prévoit que, dorénavant, la transmission des indicateurs de performance pour une année et l'application éventuelle de la majoration serait effectué non pas à l'année N plus sain, mais à l'année N plus de d'autre part, le texte prévoit le pré-remplissage de la déclaration effectuée auprès de l'Agence de l'eau avant le 1er avril ces mesures constituent de véritables simplification et sont souhaitée par toutes les parties prenantes, mais lorsque l'on parle d'eau en ce moment. Tout n'est pas aussi content il y a le problème de la compétence eau et assainissement que la loi note à faire monter obligatoirement intercommunalité a d'ici à 2020, mais il y a aussi le problème du véritable siphonage et mon collègue François Bonhomme, on a parlé du budget des agences de l'eau organisée par l'État depuis 2014 la première ponction de 210 millions d'euros devaient être exceptionnelle, elle a ensuite été fixé à 175 millions et poursuivi dans les Budgets 2015, 2016 et 2017. La voici gravé dans le marbre du PLF pour 2018 sous la forme d'un plafond morts l'État, s'autorisant à prélever des recettes dépassant le seuil de 2001 1000000000 d'euros, le prélèvement devrait atteindre un montant de 175 à 200 millions. Parallèlement, les agences de l'eau voient leurs compétences élargies au financement de l'Agence française de biodiversité pour 200 millions d'euros et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour 85 millions au total, l'État va nous ponctionner près de 460 millions aux agences de l'eau, soit 20 pourcent de de leur budget, on est bien loin du principe l'eau paye l'eau, comme l'a fait remarquer l'AMF ces prélèvements se font au détriment. Direct des collectivités puisque les agences de l'eau subventionnée projets locaux et ce, à l'heure où il faut de plus en plus mettent en oeuvre la compétence, j'ai ma pied. Il ne s'agit pas là de défendent seulement les collectivités demain les agences de l'on va-t-elle les moyens de remplir les obligations européennes en la matière, pourra-t-on satisfaire la directive cadre sur l'eau qui impose à la France d'améliorer l'état écologique de nos masses d'eau Madame la Ministre, la réponse à ces questions n'est pas des plus fluide, néanmoins le groupe UC votera cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue qui et pour terminer, la parole est à monsieur Gérard Longuet pour le groupe, les républicains, qui disposent de 2 petites minutes. Monsieur le Président, Madame le ministre et chers collègues, c'est 2 minutes ne suffiront largement car mon objectif est simplement de vous rappeler, Madame le Ministre, que le 11 janvier 2017, les présidents des 2 groupes majoritaires de du Sénat ont déposé une proposition de loi tendant ta renoncer au caractère obligatoire de la compétence eau et assainissement pour les intercommunalités, ce texte a été voté à ma connaissance et de mémoire en scrutin public, non sans scrutin public mais sans opposition, c'est-à-dire une très large majorité, correspondant à une demande très forte exprimée par les élus locaux. Le 23 février donc on en janvier : dépôt de la proposition 23 février la proposition est adoptée par le Sénat et la nouvelle assemblée, Madame le Ministre, le 12 octobre à voté un renvoi en commission. Le renvoi en commission pour une proposition parlementaire est assez rare et le sens de mon intervention. Et de savoir si vous avez l'intention, comme l'article 39 de la Constitution, vous le permet de saisir sur votre maîtrise de l'ordre du jour pour sortir de ce cette, comment pourrais-je l'a qualifié de cet emprisonnement de cette encellulement de cette proposition de loi pour la faire débattre de nouveau devant l'Assemblée, imagine très bien qu'une assemblée composée en large majorité de nouveaux élus se soit donné le temps de la réflexion réflexion pas choquant mais le temps de la réflexion sur un sujet relativement simple, a ses limites et le gouvernement à la faculté d'inscrire à l'ordre du jour, y compris une proposition de loi je souhaite savoir, madame le ministre, si c'est telle est l'intention du gouvernement, les 2 minutes sont épuisés.

Je vais répondent brièvement, monsieur le sénateur Longuet : la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles Matam a crée une compétence ciblée et obligatoires relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dites la Cette compétence, elle vise à mieux articuler l'aménagement du territoire et urbanisme avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, elle recoupe des missions d'aménagement des bassins de gestion de restauration des cours d'eau et des zones humides et et d'autres que je vais pas continuer à détailler ici la création de la compétence Jemmapes, il n'a pas donné lieu à l'attribution de missions nouvelles par rapport à celles précédemment exercé de manière partagée par tous les échelons de collectivités territoriales, la j'même qui regroupe donc au sein d'une même compétence plusieurs missions pré-existantes et l'attribue à titre obligatoire aux EPCI à fiscalité propre. Par conséquent, le mécanisme de compensation des charges transférées entre l'État et les collectivités territoriales ne s'applique pas en matière de j'aime Pour l'exercice de cette compétence une taxe facultative prévue par l'article 15 30 bis du code général des impôts est plafonnée à 40 euros par habitants résidant dans le périmètre exclusivement affecté aux dépenses liées à son exercice a été créé. Le gouvernement n'entend pas remettre en question cette compétence. et à l'article 1er je suis saisi de l'amendement numéro de rectifier, présenté par le gouvernement, Madame la Ministre. le présent amendement rédactionnel. Vise à assurer une meilleure lisibilité des dispositions prévues aux 2 premiers articles en les regroupant dans le chapitre du code de l'environnement dédié aux redevances des agences de l'eau, ceux qui sont plus approprié que le code général des collectivités territoriales.

je n'ai aucun grief au regard du fait, Madame le Ministre, que vous n'avez absolument pas répondu à ma question est qu'il y a un profond mais la malentendu il y a aucun grief donc je vote notamment mais vous n'avez pas compris parce que c'est la compétence ou et assainissement qui appartenait aux communes et qui, dans le cas de l'intercommunalité va être obligatoirement transfert mais transférer notamment aux communautés de communes qu'ils ne demandent pas, alors que nous avons des réseaux communaux parfois intercommunaux, plus petit que la connaît que la communauté de communes ou parfois plus grand que la communauté de communes qui n'ont qu'une envie, c'est de survivre et on leur demande d'adapter leur dispositif au dispositif intercommunal, ce qui l'est mécontente profondément car il part d'un principe simple : quand quelque chose marche pourquoi diable le modifier et ça n'a rien à voir avec j'Mappy j'ai parfaitement compris la politique, j'aime beaucoup plus ambitieuse, là je parle simplement d'une réalité ça fonctionne, pourquoi perturber alors que la majorité du conseil du Sénat, qui représente les collectivités locales le demande, je comprends très bien qu'une nouvelle assemblée se donne le temps de la réflexion, le temps de la réflexion doit pas durer le temps de la législature. Madame la Ministre, souhaitez vous répondre. Monsieur le sénateur, j'entends vous vous remarquez vous inquiétude et les et les questions que vous soulevez, il me semble que ce n'est pas le moment où nous devons avoir ce débat-là, vous savez comme moi que Jacqueline Gourault a annoncé un groupe de travail sur cette question-là et que ce travail va avoir lieu en concertation avec les parlementaires et les parties prenantes concernées et donc il me semble, je serai ravi et le ministre d'État également dedans, d'en parler plus en détails avec vous, mais il me semble que ce n'est pas le moment pour le faire. Merci plus d'explications de vote, je n'en vois pas donc je vois cet amendement 2 avis favorables qui vote pour. Merci, il est adopté, je suis saisi l'amendement numéro 1 présenté par le rapporteur.

de permettant, mon département d'outre-mer, le décalage de la transmission des indicateurs nécessaires à l'application éventuelle de la sanction. Monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur, le gouvernement est favorable à cet amendement car cet amendement de cohérence Viva parachever l'extension du dispositif prévu par cette proposition de loi aux offices de l'eau des départements d'outre-mer, qui avait été amorcée en commission par un amendement de monsieur le rapporteur à l'article 3 les offices de l'eau des départements d'outre-mer perçoivent également des redevances pour prélèvement pour l'eau potable et le code de l'environnement prévoit aussi un dispositif de majoration de cette redevance en cas de rendement non conforme son plan d'action, les enjeux de simplification 2 dispositifs sont les mêmes qu'en métropole

Merci, il est donc adopté mais je mais aux voir l'article 1er pas d'explications de vote. Il approuve. Je vous remercie, il est adopté à l'article 2 je suis saisi de l'amendement numéro 3 présenté par le gouvernement, M. le Ministre. Cet amendement supprime l'article 2 par cohérence avec l'amendement rédactionnel précédent du gouvernement qui importe le contenu de l'article 2 dans l'article pour

Très bien, donc je mets cet amendement doit s'il n'y a pas de demande d'explications de vote, je n'en vois pas qui approuve cet amendement. Merci, il est donc adopté et l'article est supprimé. Je mais on voit l'article 3. Pas demande explication de vote jeu mais on voit qu'ils votent pour. Merci, il est adopté l'article 4 même vote. Même vote il est adopté à l'article 5 je suis saisi l'amendement numéro 4 présenté par le gouvernement, la ministre. Monsieur le président, Mesdames, sénatrice Monsieur le Sénateur, par le présent amendement, le gouvernement entend lever le gage prévue à l'article 5 de la proposition de loi.

à l'unanimité, je vous remercie l'article est donc supprimée, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi attendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service de l'eau potable, il y a-t-il des demandes d'explications de vote.

Mais je ne vois pas d'abstention ni d'opposition, le texte est donc adopté, monsieur le président de la commission. Oui, merci Monsieur le Président, très rapidement, madame la mise mais chers collègues pour à mon tour bien sûr me me réjouir que ce texte était adopté dans cette unanimité, c'est vrai, certains ont dit que ça n'est pas un texte de grande envergure ni de grandes ambitions et c'est un texte, et Dieu sait que c'est important, très concrets, très pragmatique et qui je pense sera très et très utile aux collectivités locales, je crois qu'on y est arrivé parce que comme ça, certains l'ont dit également, on l'a fait dans dans un travail qui illustre bien, Madame la ministre, c'est que le travail sénatorial, je me permets de le dire en en adressant à vous qui connaissez moins bien cette maison que d'autres membres du gouvernement, il y a eu au départ, un travail de la délégation collectivités locales ensuite 2 co-auteur de groupes politiques différents et puis vous l'avez vu tout le monde, qui s'est rallié à cette proposition, moi, je voudrais vous remercier, Madame la Ministre d'avoir apporté le soutien de du gouvernement à ce texte et j'aimerais vous dire que je souhaite que ce soutien soit actif, c'est-à-dire que vous ouvriez de telle sorte à ce que ce texte soit rapidement inscrit à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse entrer dans les faits rapidement, juste un mot sur ce qui a été dit sur la la question du transfert de de la compétence, c'est vrai que certains ont pu avoir le le sentiment et j'avoue que j'en fais un petit peu partis que ce qu'on reprochait principalement à ce texte d'origine sénatoriale, c'était qu'il était d'origine sénatoriale, à preuve en est c'est que depuis le gouvernement a accepté de rouvrir le dossier en en en en organisant une concertation qui je l'espère, aboutira en tout cas merci encore pour votre soutien sur ce texte est vraiment, nous serions très reconnaissants qu'il soit rapidement inscrit adopté par l'Assemblée nationale merci beaucoup. Mais, chers collègues, je vous donne lecture de l'ordre du jour du mardi 31 octobre 2017 à 14 heures 30 propositions de loi attendant à soutenir les collectivités territoriales et le regroupement dans leur mission d'accueil des gens du voyage en examen conjoint avec la proposition de loi visant à renforcer les rendre plus effectives les sanctions en cas d'installation illégale en réunion sur un terrain public ou privé, à 16 heures 45 questions d'actualité au gouvernement à 17 heures 45 suite de l'examen conjoint des propositions de loi, chers collègues, Madame le ministre, la séance est levée.